L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 79 rectifier tant tendant ta inséré un article additionnel après l'article 14. oui, oui, absolument, nous allons attendre. Président de la commission rapporteur. J'ai été trop vite. Nous n'en sommes qu'aux annonces, donc tout va bien. Alors c'est. C'est

très bien, nous avons 4 amendements en discussion commune nous allons débuter. Avec l'amendement numéro 1 79 rectifier ce monsieur Laménie qui va le défendre. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, donc l'initiative de notre collègue Antoine Lefèvre et plusieurs d'entre nous, donc il est rappelé concernant cet amendement 79 rectifié, que les collectivités sont des acteurs majeurs du mécénat au bénéfice de leur territoire, les opérateurs des collectivités territoriales, telles que les SPL Les sociétés d'économie mixte contribue également à mener des actions d'intérêt général comme c'est leur rappeler dans l'objet de cet amendement et ces structures locales de petite de taille petite ou moyenne qui oeuvrent pour le compte de leurs actionnaires publics sont amenées à solliciter l'appui des entreprises privées locales pour mener à bien leur mission d'intérêt général et de rayonnement territoriale, quel est l'objet de cet amendement pour insérer un un article additionnel merci.

non, non, dans la dans la continuité avec l'objet qui exactement sensiblement le même, et pour modifier l'article 238 bis du code général des impôts, on est en en insérant année alignant comme indiqué dans l'objet de cet amendement, merci. Merci monsieur Laménie un amendement donc identique le 433 rectifier bis, il est défendu par Madame Goulet, même motif, même punition, défendu le président je vous remercie Madame Goulet. Alors quel est l'avis de la commission sur le sur ces amendements. Bonjour la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, un an, le drame avait déçu, on va pas continuer comme ça, il y aura des amendements qui nécessiteront sans doute à plus long débat donc c'est 2 amendements, nous avions déjà vu peut-être une forme un peu différente, dernière il vise à étendre le bénéfice de réductions d'impôts aux dons effectués soit aussi d'économie mixte, soit aux sociétés publiques locales agissant dans le domaine du tourisme ou de la culture, donc l'tension extrêmement louable et on comprend le intérêt d'avoir des outils qui permettent de recueillir des dons pour ce c'était ces causes qui sont par ailleurs extrêmement défendable, mais les auteurs des amendements votés pleinement satisfait parce que il est d'ores et déjà possible d'utiliser un autre type qui a été créé par la loi de modernisation de l'économie de 2008, qui sont les fonds de notation éléphants de patients peuvent comme vous le savez être créée à l'initiative de collectivités, donc une à département, une ville, une région peuvent très bien créer un fonds de agissant agissant pour le tourisme pour le Patrimoine et ce fonds est ensuite éligibles les, enfin plutôt l'aider les bébés, les donateurs à ces fonds sont ensuite lisible à réduction d'impôts donc je pense qu'il faut pas compliqué à l'envi l'édifice qui fiscaux et utiliser le véhicule qui est parti en adapté pour ça, c'est dire le fond dotation, donc c'est plutôt une invitation au retrait. Donc l'avis défavorable sur les quatre monsieur au retrait, Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. La commission a parlé d'or et le gouvernement, un avis identique. Très bien monsieur Laménie est-ce que vous retirez vos amendements. Oui, Oui, écoutez, compte tenu les explications du rapporteur général pour rester en conformité, je retire ces 2 amendements. Madame Boulet, que faites-vous identique sortirait même président Nous passons à l'examen de l'article 15. Sur cet article, nous avons 2 amendements identiques de suppression, l'amendement 236 il est défendu par Monsieur Bon, OK, pardon, Monsieur Bocquet, pardonnez-moi. Parce que ça nous arrive très souvent nous sommes voisins quasi. Bien écoutez, madame la présidente, effectivement, monsieur le ministre, chers collègues s'agit bien d'un amendement de suppression de l'article 15 ce n'est pas de l'acharnement de notre part bien compris, on est sur la taxation des transactions financières quelle bienveillance quand même de ce la part de ce gouvernement à l'endroit de la finance. Cet amendement donc alors que le Parlement a voté l'an dernier, l'élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations réalisées en une seule journée, le gouvernement entend faire marche arrière. Vous avez la constance agissant de la taxation de l'industrie financière, on l'a constaté depuis quelques jours, c'est quand même regrettable de refuser une telle taxation qui représente quand même un gain potentiel compris entre 2 et 4 milliards d'euros par an, ça n'est pas rien, alors on se souvient qu'il y a quelques semaines, sur le plan de la République avait dit à nos concitoyens guyanais qu'il n'était pas le Père Noël, en l'occurrence s'agissant là du Sri financière les cadeaux pleuvent quelques semaines de Noël c'est déjà Noël avant l'heure c'est un 1er aspect ensuite je pense que c'est aussi l'occasion de réaffirmer le primat du politique dans la gestion des affaires du monde, cette affaire-là, au-delà de l'aspect technique et budgétaire réaffirmer la puissance de l'État face établissement financier établi aujourd'hui à la City et qu'on essaie de courtiser, on assiste à des danses du ventre un peu partout en Europe, tout le monde y va de son couplet : venez chez nous vous ne paierez pas beaucoup d'impôts, on va alléger le droit du travail, c'est ce qu'on a entendu, je m'en souviens le 8 février dernier en commission des finances du Sénat dans un magnifique Consensus financier et il y avait la direction générale du Trésor il y avait, Euronext, il y avait, UBS, Morgan Stanley, le joli monde de la finance qui chantaient en choeur ce couplet : on est prêt à venir à Paris, mais s'il vous plaît, pas de taxe et alléger le droit du travail, la mission est quasiment quasiment accomplie aujourd'hui avec beaucoup de zèle par ce gouvernement, vous comprendrez dès lors le sens de cet amendement de suppression merci. Merci l'amendement 574 qui est identique, monsieur Leconte qui le défend. Merci madame la présidente, monsieur bis, mes chers collègues, oui ce qui ce qui est ce qui est dommage, c'est que finalement ce gouvernement donne l'impression de penser en silo. Parfois, il pense climat parfois ils pensait publique au développement, parfois ils pensent récupérer être attractif suite au Brexit aura l'occurrence la suppression de cet article 15, notre collègue a dit ça, répond à l'évidence, à la volonté du gouvernement d'être attractif pour le Brexit ceci étant, c'est très préoccupant par rapport à d'autres objectifs, qui sont des objectifs annoncés et des engagements du président de la République, l'engagement pour le climat, l'engagement pour monter à 0 55 euros 55 pourcent de notre revenu national, l'aide publique au développement, parce que je rappelle que ces 2 à 3 milliards qui sont prévues, qui de de rendement de de de cette taxe ont pour objectif de financer la lutte contre le choix réchauffement climatique et l'aide publique au développement, il est donc parfaitement incompréhensible que le gouvernement nous propose de supprimer 7. Taxe sur les transactions financières réalisées en une seule journée, c'était une avancée qui avait été voté par la représentation nationale précédemment et qui aujourd'hui. René finalement en cause un certain nombre d'engagements et la crédibilité du gouvernement sur des engagements en termes d'aide publique au développement et de climat, je rappelle aussi que continue de la trajectoire et de du budget du ministère Affaires étrangères il va être très difficile compte tenu de ce qui a été programmée comme baisse pour le ministère des Affaires étrangères pour les prochaines années jusqu'en 2022 de tenir les engagements du président de la République en terme de public au développement cette taxe permettait de répondre en partie à cette interrogation et ça ne pourra pas être le cas, donc nous ne comprenons pas s'être proposition du gouvernement qui, par rapport à des objectifs annoncés est absolument incompréhensible. Merci, Monsieur le comte, quel est l'avis de la commission.

les vraies difficultés de mise en oeuvre de cette taxe, je me réfère au référé la Cour des comptes, il y a un référé de la Cour des comptes que que j'ai en main dans les conclusions, je ne peux plus on a le référé de la Cour des comptes qui dressé le 19 juin 2017 au au ministre montre les importantes difficultés techniques

elle est. Plus politique, ça pénalisera évidemment à la place de Paris moi, je, je, vous savez ces taxes étaient mises en place pour la finance initiale pour 2017 nous la supprimons dès la loi de finances initiale pour 2018 ça correspond d'ailleurs totalement à une recommandation du rapport que j'ai fait sur la compétitivité de la place de Paris, après le Brexit puisque on se compare malheureusement aux autres places par rapport, notamment place allemande et le la des éléments, la compétitivité, c'est évidemment l'attractivité de la place de Paris, y compris sur le plan des, des, des taxes et des transactions et là-dessus, ça rejoint pleinement une conclusion

était un signal négatif alors ça certes vous convainc mais la 3ème raison pourrait vous convaincre, c'est chaque fois on a chaque fois on a étendu la taxe il y a eu diminution de l'assiette, voire disparition, à terme, très concrètement, si on regarde les chiffres, le rendement de la taxe était prévue initialement

les transactions ne se font plus à Paris, elles se font à l'étranger, et donc ce qui se passera ici l'estimation, on peut donner, qui est celle de l'AMF, c'est que l'extension de la taxe aux transactions intra-journalières ce. Traduirait par une diminution de 54

continueront à exister, continueront à se faire, la seule différence, c'est que ce front en dehors de la place de Paris et donc la, la, avec par ordre avec toutes les conséquences que ça représente en matière d'emploi, de fiscalité, par ailleurs, donc vous le voyez le risque et la diminution des volumes estimés à 54 pourcent, donc évidemment pour trop raison à vie et demande de retrait sinon avis défavorable. Très bien monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Merci au présidente, le gouvernement a le même avis que la Commission la taxation des opérations Intraday telle qu'avait été prévues par le la loi de finances pour 2007 est difficilement compatible avec le fonctionnement de notre TTF nationale, je rappelle que, effectivement, on a un système déclaratif Euroclear qui fait un bilan justement en fin de journée, entre les différentes opérations et que telle qu'il est paramétré et il ne peut difficilement prendre en compte l'extension que vous appelez de vos voeux, alors vous allez me dire. la France n'est pas la France, si elle n'est pas capable de mettre en place des dispositifs techniques, juridiques, etc, bon, cela étant, la Cour des comptes a quand même, comme l'a dit le rapporteur général émis un certain nombre d'observations et puis allez on assume les choses effectivement, nous ne souhaitons pas courir dans la compétition internationale avec des sabots de plomb et donc dans le cadre qui était évoqué effectivement de Brexit nous souhaitons absolument conserver l'attractivité de la place de Paris, nous nous réjouissons d'ailleurs du fait que sur la régulation, nous sommes présents et d'ailleurs si l'Autorité bancaire européenne vient à Paris, hé bien nous nous réjouissons du fait que ça ancre un peu plus je dirais l'ADN financiers de la place de Paris et pour ces raisons, nous effectivement donnant un avis défavorable à ces amendements et j'ajoute que, finalement, vous êtes en cohérence, en en proposant l'amendement du suppression de l'article et je suis en cohérence pour à l'époque n'avoir pas voté cette disposition et donc demandé le rejet de l'amendement de suppression. Très bien, Monsieur Bocquet souhaitez vous retirer cet amendement. Très bien monsieur le comte, il en est de même. oui, Monsieur le comte pour explication de vote. Oui, tout à fait la présidente, je vous remercie, je remercie le rapporteur et et Monsieur ministre de leurs explications, toutefois, elle ne me convainc pas totalement autant je suis convaincu, je suis convaincu que nous avons la responsabilité de mettre en place des taxations qui sont robustes et qui ne sont pas détournées à Blois. Donc je peux entendent sur le plan technique, l'argument sur l'assiette. mais ceci étant, je ne vois pas ici, pourquoi nous ne pourrions pas aller plus loin en la matière parce que c'est pas cet argument-là majeur qui m'a été donné l'argument majeur, c'est la l'attractivité de la place de Paris, mais l'attractivité de la place de Paris vis-à-vis de qui. Vis-à-vis d'autres capitales européennes. Alors que l'Europe est engagée, à la fois dans des démarches déclaratives, mais on attend les résultats en termes d'aide publique au développement. En termes d'accompagnement du de, de, de financement de l'accompagnement du réchauffement climatique du fond justement qui a été un

et il faudra qu'on soit attractif, alors que finalement, sur ce domaine-là, l'objectif qu'il faudrait que nous nous donnions c'est que ce type de transaction puisse être taxé de la même manière, sur l'ensemble des pays européens, le drame en la matière, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière sur le moyen et long terme, d'assurer l'attractivité de la place de Paris, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ça n'assure pas à moyen et long terme, la crédibilité de la place de Paris en terme de déclarations sur le climat ou des publique au développement. Bocquet pour explication de vote. on comprend bien l'attractivité, on comprend bien les les questions d'assiettes, on comprend bien le le référé de la Cour des comptes, mais est-ce que le gouvernement va proposer quelque chose en ce qui concerne ces ces transactions financières dont le le le sujet reste reste néanmoins entier, nous avons encore de longues journées débat et j'espère que le gouvernement pourra nous exposer sa doctrine en matière en la matière. Si merci monsieur Karoutchi pour explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, la réalité est moins sympathique que ce que l'on espère tous la dernière étude londonienne qui date de ce week-end. Ai beaucoup plus optimiste pour Londres pour Paris malgré le Brexit parce qu'en réalité les Anglais mettent en avant et c'est comme ça, au-delà du Brexit, la fiscalité, les réglementations en tous genres britannique par rapport à la fiscalité globale et aux réglementations françaises il y a pas que cette taxe, il y a tout le reste qui fait que les entreprises viennent ou ne viennent pas, alors on se montent tous au pinacle parce qu'on vient récupérer une autorité enfin pour le moment, le grand mouvement attendu de retour sur Paris des institutions financières des, des, des banques, etc, pour le moment c'est pas grand c'est pas grande rivière donc moi, je serais tenté Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, de dire qu'effectivement franchement sur cette taxe Pitié et au-delà de ça, si on veut profiter entre guillemets, j'aime pas beaucoup l'expression du Brexit il faut que le gouvernement, la région, la ville de Paris, l'ensemble des départements trouve communément des solutions d'attractivité, bien au-delà de cette taxe parce que tout y est : les transports, la réglementation, je vois que Londres veut créer carrément l'équivalent de zone franche sur la City pour dire aux gens, surtout ne partez pas, et nous nous en sommes à dire alors est-ce qu'on va changer à 0,1 pourcent Bourgogne clairement on n'est pas dans le même, on cour, ils ont compris pour garder leur truc, ils sont vraiment dans le libéralisme outrancier, c'est trop pour nous mais nous nous ne jouant que sur le fait qu'elle Brexit nous n'avons pas, je le dis de politique suffisamment dynamique alors que la région Île-de-France a créé une instance qui va directement à Londres, à la rencontre des entreprises, il faut que nous ayons une politique globale, si nous voulons faire de l'attractivité en tout cas, à Monsieur Bocquet, mais c'est pas une quelconque extension de de taxes qui va encore attirer les entreprises étrangères. Voilà, il n'y a plus d'autres demandes d'explications, monsieur le rapporteur général. Attention de de Roger Karoutchi me à l'occasion de reparler un petit peu des conséquences du Brexit et l'attractivité de la place de Paris, où il faut reconnaître que, en effet, la stratégie est un peu et le bilan, c'est un peu mitigé, donc il y a certainement une volonté qui est annoncé, il y a dans il y a dans ce PLF un certain nombre d'éléments qui vont dans le bon sens, on va parler un instant à travers la Taxe transactions financières, je pense également, on peut également penser au PLFSS je pense également, par exemple à la suppression de la dernière tranche de la taxe sur de la plus haute tranche l'attaque sur les salaires, ce sont des éléments qui vont dans le bon sens, ce qui renforce la compétitivité, notamment par rapport à Francfort, il y a également des mesures annoncées en matière de droit du travail, donc tout ça va dans le bon sens et d'ailleurs ces ces mesures regrets rejoignent les préconisations du rapport que j'ai fait sur la stratégie, pas de Brexit bon, néanmoins, tout n'est pas aussi optimiste qu'on peut l'espérer aussi est parfait que l'on peut l'annoncer pour pour 2 raisons : la première, été évoquée par Roger Karoutchi à l'instant. Nous, autant dire l'autre jour, le négociateur en chef négociateur en chef bon l'Londres restera, quelle que soit la solution passe Brixy qu'on arrive à un accord partiel qu'on arrive à aucun accord, qu'on arrive à une solution intermédiaire

de l'Europe et récupérer même carrément un certain nombre d'activités d'activités, venant notamment de l'asile et des États-Unis, grâce à un régime d'attractivité fiscale importante après sur les activités qui pourraient être perdus par Londres 10 15 20 pourcent peut-être hé bien sélectivité iront soit Francfort

qui tient moi aujourd'hui à notre fiscalité qui un mois notre droit du travail, puisque c'est aussi compliqué en Allemagne devant des licenciements qui tient peut-être un petit peu au fait de coût du travail qui reste avec les charges sociales plusieurs actifs en Allemagne mais qui tient essentiellement, essentiellement à notre image d'instabilité fiscale alors là nous supprimons une taxe va dans le bon sens, mais ces taxes a été créé la dernière et nous passons notre temps en PLF ou Opel faire à supprimer recréer des taxes qui ont été créés, recréer, donc il y a une instabilité fiscale et la France malheureusement nous avons à lutter, nous avons lutté contre City images l'orientation des choses qui vont dans le bon sens, le fait qu'on annonce une pente, une baisse de l'impôt sur les sociétés pluriannuelle, ça va dans le bon sens, le fait qu'on a un certain nombre de mesures qui soient annoncés à l'avance, tout ça va dans le bon sens, encore faut-il s'y tenir et malheureusement à chaque fois le on a eu des extensions ou des des amendements qui la dernière par exemple, ont proposé de revenir sur les régimes de cession gratuite d'actions ou des temps, la taxe comme cet effet dernière au PLF, tout cela a contribué, malheureusement à l'image de la stabilité fiscale de la France et puis partir moi la place de Paris, donc, vraiment, c'est le message que. Peut donner au gouvernement. Soyez conscient que nous sommes regardés que nous avons une image encore une fois d'un pays qui ne qui n'est pas capable de tenir ses engagements sur la durée qui est capable de défaire pas loi de finance et qui a été créé par la haute finance précédente qui est capable de modifier en paix les faits faire ce qui a été modifié, parfois 15 jours avant et donc il était important d'ici tenir nous avons soutenu samedi la baisse de la poche société avec la pente, encore faut-il s'y tenir dans le temps et je crois que c'est à ce prix que Paris regagnera de la compétitivité et de l'attractivité. Monsieur Bocquet pour explication de vote. Oui, juste une remarque, madame la présidente, je suis sur le déroulement des amendements de la science et je constate, à ma grande surprise que le 236 et 574 sont d'ores et déjà déclaré rejeté.

Absolument, monsieur le ministre, vous souhaitiez prendre la parole. Oui pour pour dire que naturellement le le gouvernement est très engagé pour créer les conditions d'une attractivité de Paris et de la France, je veux pour preuve par exemple la suppression de la dernière partie de la taxe sur les salaires, qui vise un certain nombre d'établissements justement financier pour donner un signal clair par ailleurs une mission travaille également sur des, comment dire, hé bien des des personnes qui pourraient quitter Londres non parce que leurs établissements financiers viennent à Paris, il y a un certain nombre de de demandes liées à la scolarisation par exemple un type d'éducation qu'il faut prendre en compte, il faut que nous puissions créer également ce contexte qui soit favorable et de façon plus générale vous a pas échappé que c'est l'ancien co-rapporteur du Sénat sur la loi travail qui le dit, que nous n'avons pas hésité justement à pousser les feux sur un certain nombre de tabous français et que nous sommes confiants sur le fait que ça crée un un choc favorable et en tous les cas, c'est ce que je mesure en me déplaçant près de 15 jours sur 30 à l'étranger, le regard sur notre pays change et je pense que c'est positif en termes d'attractivité voilà mais à ce stade, donc effectivement c'est toujours hé bien avis défavorables à ces amendements.

Qui est contre. Il n'est pas adoptée, il en va de même pour le 2ème amendement identique le 574 donc les 2 ne sont pas adoptées. Nous procédons à présent à l'examen de l'amendement 130 rectifier. Qui le défend Madame Boulet s'Peyronnet. Merci madame la présidente, et pardon, mes chers collègues, monsieur le Ministre, mes chers collègues, après le Brexit, donc la place de Paris à l'occasion historique de renforcer son attractivité en attirant les capitaux de la City dans la compétition fiscale qui l'oppose à l'Allemagne, la France est pénalisé par le maintien de la taxe sur les transactions financières, le présent amendement proposé par monsieur Dominati, propose en conséquence de supprimer l'article 235 terre vous du code général des impôts. Merci, quel est l'avis de la commission. La commission est tenté, puisque ça a été dit à l'instant par notre collègue, l'Allemagne et l'Allemagne et les Pays-Bas de taxe sur les transactions financières, donc évidemment c'est d'Avantage compétitif pour eux est défavorable pour la France pourrait tout à fait complet si l'on parle de Londres Le Royaume-Uni à une taxe qui est un droit de timbre dont le rendement est de lors 2 un milliard de livres donc à peu près équivalent à ce que nous donne un peu moins que le rendement de d'attaque, ce qui est d'un milliard 5 pour la France, donc évidemment ça serait si on voulait aller jusqu'au bout la logique tout à fait normal, normal, logique de supprimer totalement la taxe, mais c'est une perte de recettes de 1 milliard 5, dont plus de la moitié des recettes affectées au fond de sa vérité pour le développement, il y a aussi des collègues qui sont d'ailleurs dans la commission des finances, rapporteur qui nous ont dit la la difficulté qu'il y avait pour abonder les fonds chargé en matière de développement, à un moment où je pense que la question de l'immigration, notamment l'immigration illégale en Europe se pose et où l'aide au développement ne doit pas être relâchés donc pour ces raisons, et au grand regret qu'on peut avoir grand coup peut avoir quant à la compétitivité, la place de Paris, c'est une demande de retrait continue la perte de recettes et compte tenu de la difficulté de retrouver des ressources pour le développement, donc, pour ces raisons vendredi. l'avis du gouvernement. convergence effectivement fiscales notamment et et social et donc notre idée, c'est en prenant appui sur la la TTF française nationale, hé bien de, de, de créer une TTF européenne, c'est ce qu'il a indiqué dans dans son discours de la Sorbonne, et par ailleurs effectivement comme l'a souligné le le rapporteur général, la perte de recettes et de un milliard 5 alors je sais que la semaine dernière un PLFSS a été voté avec je crois 7 milliards d'euros de différentiel mais bon, pour autant, il est compliqué de donc de faire aboutir votre proposition mais je reconnais là, hé bien, en tous les cas, la persévérance de Philippe Dominati et la vôtre effectivement dans le sens de plus de liberté, mais en même temps, voilà en même temps il faut il faut également avoir des outils permettant de de financer une politique ambitieuse d'aide au développement je peut-être à l'occasion d'y revenir un peu plus tard mais donc c'est une demande de retrait à ce stade, rejet. Madame vous Boulez Peroni est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement. Oui, j'ai bien de quel côté constructif de la réponse du rapporteur général du Ministre je montre le lien, sans jeu de mots fallacieux en retirant l'amendement. Mon nom est retirée. Nous procédons à présent à l'examen de 2 amendements identiques, le 237 il est défendu par monsieur Oui, cette amendement visant à donc remonter le taux de prélèvement de la taxe sur les transactions financières de 0 3 à 0 5 ce qui est quand même pas une approche maximaliste. C'est dégagé des nouvelles recettes pour l'État et dans le cas des engagements pris par la France en matière d'aide au développement et on va rebondir sur le débat que nous avons eues précédemment. En effet, ça fait presque 50 ans que notre pays, comme tous les pays de l'OCDE a pris l'engagement, dans une résolution de l'ONU de consacrer 0 7 pourcent de son PIB à la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique, d'une part et le soutien au développement de la solidarité internationale et l'amélioration de la santé mondiale ce seuil ne vient pas de nulle part, il a été déterminé par le prix Nobel d'économie qui voit le seuil permettant aux pays émergents de connaître un développement durable et indépendant, au final, si on pourrait dire que si on continue à le non-respect de ce seuil, l'aide publique au développement est voit à disparaître, c'était que cet engagement, certains pays l'ont respecté et ce dès 1975 tout à l'heure on on voyageait a été à Londres, on va revenir peut-être en Allemagne, dans nos débats, ben je vais citer moi le Danemark, la Suède, la Norvège et là on peut pas m'accuser, je vais même citer les très libéraux des Royaume-Uni et du Luxembourg ou encore le modèle qui vient souvent souvent vanté dans nos échanges, l'Allemagne, tous l'ont fait. Tout ce l'on fait. On pourrait y ajouter et manque de pot pour mes collègues ont même maintenant, les États-Unis vont. En matière d'investissement rapide en matière d'aide au développement, alors c'est pas par philanthropie c'est pas par alignement zélé sur les résolutions de l'ONU, c'est parce que tous les pays développés ont un certain intérêt à s'engager dans le développement des pays émergents. Parce que les Liens entre pauvreté conflits armés et terrorisme fait est, en fait, depuis plusieurs décennies, parce que nous sommes dans un monde globalisé et que la pauvreté là-bas produit toujours des troubles ici parce que, qu'économiquement les pays émergents sont un formidable vivier de main-d'Oeuvres et de partenariats commerciaux, comme le rappelait le G8 en 2005, je finis encore sur les Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ont, ils ont su trouver un essor dans la société civile, mais aussi dans des structures étatiques, Forte pour développer leurs réseaux et leurs investissements, donc nous parlons de la nation et son rayonnement là. Pour donner qu'un chiffre, l'Agence de coopération internationale allemande la guise compte 17000 employées et concentre plus de 2 milliards d'euros de dotation, Monsieur le Ministre, c'est le double. En termes d'investissements par rapport à notre Agence française de développement et le décuple en terme de salariés notre AFD donc vraiment montons un peu ce taux de 0 3 à 0 5 pour que la France retrouve sa place au niveau international, merci. Sur l'amendement 322 rectifier qui est identique, c'est Monsieur le qui le défend. Oui, tout à fait, merci madame la présidente, monsieur Miss, mes chers collègues, je salue l'argumentation de notre rapporteur, il nous explique pourquoi effectivement il faut maintenir cette taxe et maintenant encore plus, le Sénat a suivi les les propositions du gouvernement, qui consistait à à finalement réduire l'assiette pour que ce soit plus robuste, alors pourquoi ne pas remonter un peu ce qu'il reste de la taxe sur les transactions financières pour essayer d'accompagner notre objectif de monter à 0 55 pourcent du PIB pour les publics au développement,

à nous handicapés et à ne pas nous permettent de développer un certain nombre de politiques, qui sont pourtant annoncée, je m'interroge sur l'intérêt de cette activité cette attractivité, elle doit dans une utilité, l'utilité, c'est justement de pouvoir avoir plus de moyens pour développer des politiques et pas le contraire, alors là au nom de l'attractivité en fait on se on on abandonne la notre capacité de développer des politiques eux-mêmes, notre partenaire, les plus libéraux mettent en oeuvre de manière plus efficace. Quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements. Pour entendre ce que l'on dit sur Luxembourg sur l'Allemagne sur le Royaume-Uni, qui apporterait une aide médias des dépenses supérieures à celle de la France, le seul problème c'est que votre amendement ne résout absolument rien puisqu'il y a plafonnement des ressources de l'AFD, donc vous pouvez remonter le taux le quintuplé comme vous faites ça ne se produirait strictement rien en terme de ressources pour l'Agence française de développement du fait du plafonnement donc malheureusement ça c'est par contre ça aurait des effets assez catastrophique sur l'attractivité de la place de Paris puisque les pays que vous avez cité par ailleurs, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, par exemple, n'ont pas de taxes transactions financières donc la la France, on aura une Elsa quintuplé, donc vous imaginez les le, le risque c'est évidemment que l'assiette disparaissent puisque les capitaux sont mobiles, il n'y aura plus de transactions de ce type en France et en revanche il y en aura en Allemagne il y un arrêt aux Pays-Bas il y en a, Luxembourg, qui tous ces pays n'ont pas de transaction transactions financières, non mais oui, mais, mais dans la pratique, Camilla plafonnement des ressources de l'AFD Trabant votre amendement comme un plafonnement des ressources de l'vider votre plafonnement est sans effet sur les ressources de l'AFD donc malheureusement avis défavorable. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente, alors vous le savez, monsieur sénateur le le taux initialement prévu lors de la création de la TTF a déjà été triplé. D'ailleurs, on est passé l'année dernière. En 2017 de 0 2 à 0 3 pourcent et on n'a pas encore d'ailleurs pu appréhender l'ensemble des effets de cette hausse et si le Royaume-Uni que vous évoquiez, on est à 0 5 pourcent il faut voir que la législation britannique prévoit un grand nombre d'exonérations, comme par hasard, sans commune mesure avec celles qui existent en France et que du coup, en fait, échappent à la taxe là-bas, en dépit de son toit 05 toutes les activités financières des banques de financement et d'investissement, là où la taxe foncière française n'exonère que les activités liées à la tenue de marché, donc pour nous, il faut en rester là et puis puisque était évoqué effectivement la politique française de développement, pardon de dire que le précédent quinquennat c'est pas eu. En la matière, prenez la courbe, prenez la courbe pour le coup, elle s'est inversée, là véritablement et donc

Jean-Yves Le Drian et votre serviteur travaille d'ailleurs à une nouvelle courbe pourquoi ce ce que cela soit pris en compte par nos amis de Bercy, j'en profite ce que j'ai le micro commis d'office. Je peux prendre des engagements de ce point de vue-là qui pourront s'appliquer, mais. Chef de plaisanterie, nous nous y travaillons pour avoir véritablement une ambition effectivement faire en sorte que la France soit à la hauteur de son ambition de ce point de vue-là mais donc, à ce stade et pour les raisons d'ailleurs qui évoquait le rapporteur général, c'est une demande de retrait, c'est mon avis défavorable. Monsieur Karoutchi pour explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je je comprends très bien qu'on dise, l'aide au développement est très faible, trop faible, mais pardon de vous le rappeler que avant l'existence avant la création de cette taxe, l'aide au développement était beaucoup plus forte, donc je vois pas très bien pourquoi on veut absolument sinon sur les ressources de l'AFD lier les 2, trouvons des éléments de politique en interne permettant d'accroître l'aide au développement, il une réelle politique d'aide au développement, mais ne faisons pas de la taxation financière, la seule ressource de l'aide au développement, sinon par définition vous allez empêcher les entreprises quelles qu'elles soient de venir s'installer, donc vous aurez moins de ressources, moins de ressources, moins de capacité à faire de l'aide au développement, bien il faut pas que ce soit un système où finalement tout le monde est perdant et vous n'aiderait pas l'aide au développement, juste une remarque, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur du temps glorieux Augereau présenté la France auprès de l'OCDE, j'ai essayé d'obtenir au moins une chose que je n'ai pas obtenu, je vous rassure tout de suite, à savoir d'avoir la même définition. Du taux de l'aide des des différents États dans l'aide au développement, parce que quand on regarde bien, Alain ce que ce que chacun des États, mais à l'intérieur de l'aide au développement, on n'a pas du tout la même chose, mais alors pas du tout la même chose, certains intègrent leurs territoires ultramarins, d'autres ne les intègrent pas certains intègrent des aides qui ne sont en réalité à pas des aides publiques, donc il faudrait avoir déjà les mêmes critères, les mêmes définitions comparer, ça n'empêche que ce qui est vrai c'est que l'aide au développement française affaiblie qu'on peut, on doit l'augmenter, mais ne faisons pas un lien avec la taxe financière. Monsieur Dallier pour explication de vote. Merci madame la présidente, monsieur mini-semi-chers collègues mon intervention dans le même sens que celle de Roger Karoutchi, si nous souhaitons augmenter le niveau de la de développement en France, mais faisons-le directement sur le budget de l'État, faudrait-il encore s'en donner les moyens, alors c'est vrai, quand on a le mal quand on est en Allemagne, avec un excédent budgétaire de 20 ou 30 milliards, c'est plus facile que quand on est ici, avec un déficit qui va dépasser les 80 milliards mais vouloir utiliser des affects, des des taxes affectées, on voit effectivement à la limite de l'exercice, pourquoi les pénaliser un secteur pour aller infecter une taxe alors certes une belle cause c'est un peu la même chose avec le l'impact sur les les billets d'avion, alors certes les financer la lutte contre le SIDA, ou aller financer l'aide au développement, c'est très bien mais on cible particulièrement un secteur et puis après on s'étonne que dans le secteur bancaire, les banques irais choisir une autre place que la place de Paris, mais il faut être absolument logique donc, mes chers collègues, j'allais, j'ai envie dire n'en rajoutons pas et pour répondre à monsieur Leconte je dois dire que John Reid je ne regrette pas d'être venu ce matin de bonheur parce que j'ai enfin compris pourquoi l'jamais tomber d'accord, vous vous parlez dumping fiscal, quand il s'agit pour nous de nous remettre à peu près dans la moyenne européenne, c'est quand même extraordinaire, vous pourriez nous qualifier effectivement qualifié ce que nous faisons ce que fait le gouvernement actuellement de Billy Crystal si on essayait de se mettre au niveau de l'Irlande ou d'un certain nombre de pays et vous êtes utilisé le même terme alors que nous sommes très au-dessus de la moyenne et qu'on essaie de revenir dans la moyenne, donc on n'arrivera jamais à se comprendre, je ne regrette pas d'être venu ce matin.

L'explosion de la finance constatée depuis des décennies peut-être le le l'interview de du prix Nobel d'économie, Mohamed Yunus il y a quelque temps, et on l'interrogeait pour savoir si, 10 ans après la crise financière, les leçons avaient été tirées il répond ceci n'ont aucune au lieu de saisir l'occasion de repenser le système, on est reparti comme avant, trop content de s'être réveillé d'un long cauchemar, pourtant, nous sommes toujours dans une crise liée à la concentration des richesses favorisée par le capitalisme aujourd'hui sur la planète 8 personnes détiennent davantage que 50 pourcent des moins riches, soit 4 milliards d'individus, c'est pas du discours de propagande, c'est une réalité, c'est 8 personnes, ils étaient 58 en 2015 les mettait à l'époque dans un bus Macron et ils étaient en 2010 388 on les mettait dans un Airbus maintenant, ils sont 8, c'est une petite voiturette de golf, voyez, et demain dans 25 ans, à ce rythme d'évolution là il y aura dans le monde, le 1er trilliards air du monde dont la fortune s'estimera en milliers de milliards aurait 25 ans pour les dépenser en raison des dépenses d'un 1000000 de dollars par jour, voilà où nous en sommes, vous êtes d'accord avec ça ou pas, voilà la question que l'on pose au-delà la taxation où va ce système vous allez nourrir la finance folle dérégulée qui va enfler et un jour exploser et peut-être pendant très longtemps.

de programmation des finances publiques relatifs au relatives au crédit du ministère et affaires étrangères donc aussi les publique au développement 2018, 2,86 milliards 2019, 2 75 milliards 2020, 2,66 milliards, c'est ce que le gouvernement nous a proposé comme trajectoire des finances publiques, donc si au niveau au bord du gouvernement et dans la majorité de cette assemblée, nous sommes d'accord pour dire oui, il faut faire des efforts et donc cette trajectoire n'est pas acceptable, il en faut une autre et qui a une majorité pour ça et que le gouvernement s'engage, comme vous l'avez indiqué ce matin, alors ce débat a déjà eu du bon, deuxièmement, je pense que, effectivement, on peut si on est dans des jeux de rôle, on ne se comprend pas, je n'ai pas dit ça, non, je n'ai pas dit ça, de cette manière-là, ce que je n'accepte pas, c'est l'argument qui consiste à dire que puisque nous devons être attractifs. Nous devons finalement développer un certain nombre de politiques pour que les banques qui sont aujourd'hui à Londres viennent chez nous, plutôt qu'à Francfort ou à Madrid. Oui, mais c'est sur les bancs du rapporteur et du gouvernement, que j'ai entendu ces arguments, moi je, je, je ne mets pas que quand on explique l'attractivité de la place de Paris, elle doit pas c'est pas l'attractivité de la place de Paris par rapport à Singapour, c'est l'attractivité de la place de Paris par rapport à d'autres capitales européennes et qui doivent être effectivement toute réguler les avec les vôtres et puis vous savez, je 2 de ce point de vue là je crois que alors on on voit ce que veut dire l'explosion de la finance, l'explosion des engagements, l'explosion des engagements des banques par rapport à l'économie réelle, nous avons déjà vécu ça en 2008, nous avons vu ce que ça veut dire. Et nous ne pouvons pas sous prétexte que tout va un peu mieux aujourd'hui en terme de de financer cette perspective de croissance, se dire reprenons tout de la même manière qu'en 2008 non, le problème majeur, c'est que tant si on encourage une poursuite par les produits dérivés, par un certain nombre de choses du décalage qu'il peut y avoir entre l'économie réelle et la croissance des engagements financiers des opérateurs financiers, nous sommes de plus en plus fragile. Voilà et on ne peut pas rester dans cette dynamique-là. Monsieur rapporteur général. On peut tous s'entendent sur le fait que la France peut et j'évoquais le contexte international, à la question de malheureusement d'immigration et elle avait dit ici la difficulté que nous avons la réguler, et on peut tous s'entendent sur la nécessité d'avoir évidemment un budget pour les développements plus important, la seule difficulté, c'est que cet amendement ne résout strictement rien, il y a plafonnement. Des ressources de l'AFD, donc c'est vraiment de la pétition de pure forme, pouvez-vous dire quintupler la taxe, comme vous le faites, vous n'aurez pas un centime de plus pour l'AFD, donc c'est la première, première chose, deuxièmement je le dit : si vous avez cité sainte de pays, tous ces pays, l'exception de l'Angleterre qui a un droit de timbre, non pas de taxer les transactions financières, donc la conclusion, elle est celle qui a été évoqué par certains, la taxe n'a de pertinence que si elle s'instaure dans un cadre européen, sinon il y a des placements instantanée des capitaux, j'entends ce que dit Éric Bocquet que la finance est folle que on arrive à des trillions etc Bordeaux tout ça simplement voilà, nous ne sommes pas isolé sur une plaie, nous sommes pas seuls sur la planète, rien ne bouge plus que les capitaux et si la France est le seul pays à avoir des taxes, à niveau élevé, hé bien ce sera le seul pays où les capitaux Fillon voilà, c'est tout simplement ça, donc s'il y a des propositions d'extension de la taxe au niveau européen, on peut y souscrire mais être les seuls à vouloir apporter la vertu pour le monde entier a été le seul à vouloir taxer, hé bien nous serons les seuls à ne plus avoir de place financière, ce sera le début de la conclusion auquel iront les investisseurs, c'est ce qui s'est passé, chaque fois, chaque fois on est étendu la base le rendement a baissé, voilà donc il y a une auto-destruction de la base, il y a une corrélation directe sur l'augmentation du taux et la diminution de ressources malheureusement les capitaux vont ailleurs, et on le voit chaque fois. Madame Keller pour explication de vote. Merci madame la présidente, je voudrais soutenir les termes de l'explication à l'instant du rapporteur général, nous faisons tout ce constat que l'aide publique au développement française est insuffisante, l'étalement la moitié de ce que finance Allemagne ou le Royaume-Uni, malgré la dette importante historique du Royaume-Uni, donc c'est la question du Consensus naziunale autour de cette priorité du développement et l'augmentation de la TTF techniquement n'a pas d'effet à cause du plafonnement des ressources de la FED, qui pourtant conduit des projets importants et stratégiques dans les pays du Sud, je voudrais en témoigner en tant qu'ancienne, administrateur de la deuxièmement, je crois qu'il faut regarder cette TTF en face, ce n'est pas un impôt qui va limiter le développement à l'excès des produits structurés malheureusement chers collègues pour un tas de raisons techniques, c'est un impôt de bourse qui est applicable au produit produit dont on connaît l'existence, donc ça n'a pas d'effet que vous appelez de vos voeux sur des transactions qui serait dangereuse et comme l'a dit très clairement, le rapporteur général, le bon niveau c'est effectivement européen voire OCDE hein, de manière à ce que si un instrument financier mis en place, il soit très largement partagé, enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais souligner l'engagement de votre gouvernement, sur le fond, c'est-à-dire l'aide publique au développement, on a tous conscience que sur les décennies à venir, l'enjeu des pays du sud de la démographie, de la montée de la pauvreté est majeur : le l'orientation, vous donnez à ses têtes publique au développement, va dans le bon sens mais à charge pour nous aussi de développer un consensus sur le fait que des moyens budgétaires significatifs en progression doivent lui être accordé, je vous remercie. Sur le 237 qui est pour, avec 2 pardon avec 2 avis défavorables 237 ce qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adoptée, il en va de même pour le 322. le 322. Sur l'article 15 il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Je n'en vois pas qui est pour. qui est pour. L'article 15 être adopté. Article additionnel après l'article 15 nous avons un amendement 265 rectifier terre. C'est Madame Madame Di Folco qui le défend. Merci madame la présidente, cet amendement est inspirée de la proposition de loi tendant à faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce qui a été enregistrée le 2 mars dernier il vise à mettre fin au moment du divorce à la taxation de l'attribution d'un bien propre de l'un des époux à l'autre époux en paiement d'une prestation compensatoire en capital, en effet, l'administration fiscale considère que cette attribution doit être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-values immobilières imposables cette interprétation a pour conséquence de rendre peu attractifs, ce mode de règlement de la prestation compensatoire, en ajoutant à cette opération, une imposition supplémentaire absente des autres modalités de versement merci. de la commission. Collègues c'est amendement c'est la traduction de la proposition de loi qui porte le numéro 449 sur les conséquences pécuniaires du divorce en exonérant de plus-Value immobilière les biens attribués à type de prestation compensatoire bon le coup a semblé assez limitée à la Commission, donc, c'était pour il y a une vision plutôt bienveillant de cet amendement parce qu'on comprend évidemment que c'est traité comme une plus-Value, ça n'a pas partir mandataire d'avoir aidé des biens attribués a été de compenser une prestation compensatoire, néanmoins, n'ayant pas pu expertiser l'impact sur les finances publiques, la commission souhaite entend le garnement sur cet amendement. Quel est l'avis du gouvernement. en 2014 je me réfère à ce que disait le rapporteur général, il y a quelques instants, la nécessité aussi d'avoir une certaine stabilité fiscale, de ne pas faire évoluer les les régimes chaque année et donc pour la pour nous c'est un effectivement une demande de retrait, on a, on n'a pas de dévaluation robuste du coût de la mesure, à ce stade, et par ailleurs effectivement lorsque les réaliser cette cession en exécution du décision de justice le le droit véritablement que ce soit soumis à l'imposition des plus values Molière mais surtout je crois que c'est l'argument de de stabilité, nonobstant le fait que voilà, il peut y avoir des cas ici ou là qui doit pour nous l'emporter, donc c'est une demande de retrait de la présidente. Madame Goulet pour explication de vote. Madame la présidente, monsieur ministre, mes chers collègues, l'amendement de notre collègue qui est quand même frappé au coin du bon sens, c'est pas, c'est pas une session n'importe laquelle, c'est une session dans le cas d'un d'un divorce, il est tout à fait logique, on a plutôt intérêt en la matière à à procéder par voie de prestation compensatoire, mais que la taxation qui y vient afférentes ne ne rend pas attractif ce mode de règlement qui est pourtant qui est pourtant souhaitée, donc on n'est pas dans ce, dans le cas d'une cession n'est pas dans le cas d'une instabilité on est juste dans le cas d'un règlement thématique dans le cas de session, il y a une prestation compensatoire, dans le cas d'un divorce, donc chacun reconnaîtra que c'était une modalité un peu particulières, et que ça n'a rien à voir avec une instabilité législative ou fiscale, donc moi je soutiendrai l'amendement de François Pillet. Madame Prima pour explication de vote. des du du travail législatif que nous menons ici arriver que nous lui laissions passer une forme d'injustice entre différents régimes, donc je pense que là il s'agit d'un correctif pour rétablir une injustice dans le cadre particulier, d'un d'un divorce qui n'est pas l'essence même de la transaction financière, donc je pense qu'en tout cas moi je soutiendrai cet amendement. Il y a-t-il d'autre demande explication de vote Monsieur le ministre. Ce qui est bien dans cette période c'est qu'on a l'occasion de se revoir régulièrement entre la discussion du PLF la discussion des collectifs et donc moi ce que j'aurais tendance à vous proposer en méthode c'est pour qu'on puisse faire du bon travail, c'est se donner quelques jours puisque le PLFR viendra vient devant l'Assemblée la semaine prochaine, viendra ensuite ici sur quelques jours pour avoir une vision un peu plus complète des coûts en question et, par ailleurs, voilà,

Madame Di Folco est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement. Côté contenu de du regard bienveillant de la commission et monsieur le rapporteur général et du soutien de mes collègues, je maintiens l'amendement. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement. La Commission demander l'avis du gouvernement, le gouvernement a proposé un retrait qui est pour. qui est pour. L'amendement était adopté. L'amendement 434 rectifier. Il est défendu par. Madame Goulet peut-être Madame Loisy ou Madame Sempé alors Madame Goulet. Voilà, pardonnez moi j'étais sur la sur l'amendement précédent, il s'agit dans cet amendement de réformer les plus-values de cessions immobilières encore. Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en fait valorisant les détentions longues juridiquement ça se manifeste par un taux d'imposition de 19 pourcent un taux de prélèvement social de 15 et demi pour 100 et un double régime d'abattement fiscal et social, selon la durée de la détention, cette double finalité a eu son utilité, sa justification économique toutefois ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la crise du logement et la crise de la construction dont souffre une large partie de la population, c'est au bénéfice de ses observations qui est présentée ce présente amendements dont le 1er cosignataires et Vincent de La chaux merci. Chers collègues, quel est l'avis de la commission. En commission, il avait été suggéré de Vincent Delay de retirer l'amendement pour le redéposer en 2ème parce qu'on est parti dans la mesure où très concrètement, il prévoit une entrée en vigueur au 31 décembre 2016

que d'avoir des simulations et il y a un impact financier de la mesure de la part du gouvernement et Vincent Delerm, lorsque nous avons examiné certes brièvement ce que nous avons examiné s'amendement en commission avait indiqué qu'il leur retirait pour un examen en seconde partie, donc je pense que les télés sera d'accord. L'avis du gouvernement. C'est exactement le même avis de méthode, hein, que la commission. Madame Goulet est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement oui. Défaillance de la transmission, madame la présidente, il est retiré. Il est retiré. Nous examinons à présent l'amendement 394 rectifier c'est Monsieur Bocquet qui le dit. pour répliquer à remarque de notre collègue Fabienne Keller et rapporteur général très respectueusement effectivement au niveau européen, c'est l'effet échelon pertinent, on est d'accord pour l'application de cette taxe, le problème c'est que ce gouvernement, on peut s'interroger savent volonté politique de faire les choses puisque monsieur Macron à peine élu, le lundi 22 mai demander le report d'une réunion prévue en marge de l'Eurogroupe, qui était l'occasion d'aboutir à un accord entre les 11 pays européens constituer en coopération renforcée depuis 2011 suite à l'impossibilité de trouver un accord avec tous les États membres de l'Union européenne, mais Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sur les économies ont préféré la reporter, où est la volonté politique de ce gouvernement. Quel est l'avis de la commission. Le débat a déjà eu lieu, donc vous courez que la vie soit défavorable, ensuite, on peut avoir tué un argumentaire sur l'utilité pour les teneurs de marché d'État d'avoir un marché fluide, c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui une exonération donc avis défavorable. Et du gouvernement. Oui, même avis effectivement les activités de de tenue de marché ont pour objet d'apporter de la liquidité au marché de limiter la volatilité volatilité des cours, donc voilà sans activités qui sont importantes et leur exonération apparaît justifié comme le sous-entendait à l'instant, le rapporteur général, donc avis défavorable. Y a-t-il des demandes, explications de vote. Je n'en vois pas je vais mettre au voile, amendement 394 rectifier assorti de 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adoptée. Nous allons examiner l'amendement 395. Monsieur Merci madame la présidente, donc Monsieur le Ministre, mais mes chers collègues, l'on est dans le même esprit que l'amendement précédent puisqu'il s'agit ici de mettre à contribution les les remarquables investisseurs qui souscrivent les femmes. Crédit défaut soit absous comptera sur défaut de crédit. Je vais pas ici vous décrire le le le processus par lequel les souscripteurs de tels produits dégagent des profits, mais c'est de manière obligé sur le dos des débiteurs les plus faibles. On sait que de tels contrats avaient été souscrits à l'époque de l'émergence de la dette publique grecque et que l'espérance de gain de cette nature ne semble pas avoir abandonné les acteurs des marchés financiers, nous avons raison d'ailleurs de, de, de nous inviter dans le débat sur l'Europe, on le fait régulièrement ici, nous ne sommes plus évidemment dans la période des années 2008 2009. Ou la thrombose des marchés financiers nés de la crise immobilière états-unienne avait provoqué quand même une flambée. Des assurances de prêts à hauteur de 60000 milliards de dollars. Mais le stock de contrats de cesse assurance de prêt aujourd'hui estimé à 12000 milliards de dollars et qu'il peut connaître ces prochaines années, une forme de relance pour peu que la crise systémique du secteur bancaire italien ne trouve guère d'autre issue que celle de la fermeture de plusieurs établissements ou que la bulle de la dette, étudiante américaine ne se diffuse en produits dérivés ou des produits hybrides, sans parler de la dette publique grecque toujours contenu dans les écritures du mécanisme européen de solidarité

donc, vous savez que la dernière si vous souvenez bien, nous avions d'ailleurs proposé de toiletter le code général des impôts et supprimer pour être très précis : l'article 235 Ted Tairraz aidé du choléra des impôts puisque il vise une taxe qui. à rendement 0 parce qu'il porte sur une assiette qui est elle-même interdite par le règlement européen, donc tout ça et l'appui du pur affichage donc la bon le grondement s'étaient opposés pour des raisons symboliques, mais comme il y a pas de au regard de notre l'argumentation européenne il n'y a pas de rendement, donc on peut la quintuplé et je peux même vous donner un avis favorable sur 1000 pourcent ça rapportera toujours 0 donc merci avis défavorable. Oui, même avis que la Commission et et d'ailleurs je crois qu'on peut, du coup, à réfléchir à la suppression pure et simple, un dispositif qui est purement virtuelle, voilà, donc je crois que le travail va être engagée entre la Commission, le gouvernement de ce qu'on a vu là, pour les prochaines échéances budgétaires. y a-t-il des demandes d'explications de vote Monsieur Savoldelli. La première, ça serait bien qu'on est un peu plus d'éclairage, monsieur le ministre, du point de vue du de ce que va être l'attitude de la France au sein de l'Europe. On mérite quand même ici quelque soient nos analyses, de, de, d'avoir un cap quand même un peu plus précis quand on regarde la succession des amendements. Premières remarques et 2 par esprit de responsabilité, nous retirons l'amendement. L'amendement 395 et retiré, nous examinons à présent l'amendement 306 rectifier bis c'est Madame Loisy et qui va le défendre. Merci madame la présidente, machinisme, chers collègues, l'objet de cet amendement à recettes égale pour l'État, c'est d'adapter les prélèvements fiscaux à la réalité économique pour les paris hippiques, sportifs et Poker en fondant la fiscalité sur le produit brut des jeux, le PDJ est constitué des enjeux moins le retour parieurs, c'est-à-dire y compris tout montant donné aux parieurs, le PDJ constitue donc le véritable revenu des opérateurs de paris le passage au prélèvement sur le PBJ permettrait aux opérateurs et à l'État un partage de sort, ce qui ne remet pas en cause une taxation sur les enjeux qui représente, je le dis, le volume d'activité et non le revenu concernant le pari hippique, qui fait vivre, je le rappelle toute une filière et représente plus de 80000 emplois non délocalisables, il serait ainsi envisageable de relever progressivement le taux de retour parieurs pour redonner ainsi une attractivité au Paris ces dernières années plusieurs rapports ont souligné l'effet contraignant du prélèvement sur l'mises des joueurs et non sur le PBJ qui je rappelle est opérationnel jusqu'en 2010, l'Arjel notamment a noté dans son rapport que l'assiette sur les Miss se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché, les opérateurs sont imposées sur des sommes donc qui ne perçoivent pas de la commune, la Cour des comptes en 2016 confirme également que la fiscalité française est lourde en raison de ses choix d'assiette sur les mises, d'autant que les taux sont élevés et, dernièrement, un rapport de l'Assemblée nationale, estimait qu'il était contestable de continuer à adopter comme assiette les milices qui ne font que transiter chez l'opérateur, cet amendement propose donc de modifier les taux des prélèvements pour tenir compte de ce changement d'assiette les niveaux proposés assure la neutralité de l'amendement pour les recettes fiscales de l'État, des opérateurs de la sécurité sociale et des collectivités locales les changements induits pourraient profiter assez rapidement à l'État qui consoliderait ainsi une source de recettes et enfin je le rappelle, un véritable levier pour relancer les paris hippiques du PMU et les recettes de toute la filière, merci.

dans le temps qui était imparti à la commission, nous n'avons pas pu mesurer l'impact de cet amendement, qui est assez significatif, je disais qui, par ailleurs, vous savez qu'il y a une affectation d'une partie du produit au sommet, celle du sport ne modifierait pas les ressources du certes déjà du sport puisque de façon il y a plafonnement mais je le dis clairement la difficulté a été d'expertiser les conséquences de cet amendement assez technique assez long et c'est la raison pour laquelle la Commission avant de se prononcer, soit le gouvernement, sur cet amendement. Eh bien, quel est l'avis du gouvernement. notamment la filière équine et donc. Je comprends qu'elle souhaite donner une attractivité meilleur un certain nombre d'outils liés au jeu, cela étant, nous sommes comme la commission et le gouvernement, nonobstant le fait que une capacité d'expertise dans un service importante, nous n'avons pas pu non plus avoir une étude d'impact suffisamment solide, parce que le le la modification vous proposez, elle est, elle est substantiel puisque effectivement désormais la la fiscalité ne serait puis assise sur les mises des joueurs, mais sur le produit brut donc défalquer effectivement du paiement des des gagnants, par ailleurs, l'amendement aurait aussi comme conséquence, un monde de la fiscalité sur les opérateurs en ligne qui sont majoritairement basés à l'étranger notamment à Malte et donc moi je pense que il serait de bonne politique en tous les cas que le ministère du du budget et faire des comptes publics un rôle important par rapport à un certain nombre d'opérateurs du secteur puisse utilement travailler avec vous, là aussi, afin de déjouer de calibrer de voir les mesures qui pourraient être utilement prise pour conforter ses ces filières qui dans nos territoire vous vous évoquiez le PMU naturellement finance permet de financer des secteurs importants mais, encore une fois, c'est pas une petite affaire le gouvernement, à ce stade. Du coup, et même une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable. Madame Loisy est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement. Non j'ai pas de retirer, président, ce que je, je, j'insiste sur le fait que les taux qui sont proposés ont tenu compte en fait du changement d'assiette et s'inscrivent dans une perspective de neutralité, alors je comprends, il n'y a peut-être pas eu suffisamment de temps pour analyser toutes les retombées, néanmoins je, je, je pense que le fondement de cet article est bon et et que ça ne durera pas une baisse de la fiscalité pour les les opérateurs étrangers puisque, une fois de plus, les, les, les taux seront revalorisées voilà donc moi je, je maintiens certains moments parce que l'enjeu pour la filière est et on n'a pas encore une année. De année. De lèche pour explication de vote. Merci madame la présidente, moi je voterai cet amendement pourquoi j'entends bien, Monsieur le Ministre, vous nous dites, on est prêt à étudier, à Bercy, mais tous les ans on a déjà eu le coup avec la TVA européenne, Bercy était prêt, la Bercy est encore prêt moi je voudrais insister sur le fait que la filière hippique qui trouve une part de son financement au travers du pays, ce sont des vrais emplois, c'est ce que vous appelez de l'économie réelle, c'est de l'aménagement du territoire, donc pour toutes ces raisons, moi je remercie Madame Losier d'avoir déposé cet amendement pour que le débat soit effectivement ouvert et je pense que le meilleur moyen d'ouvrir le débat, c'est de voter l'amendement ça permettra à Bercy pour une fois, de ne pas attendent l'année prochaine en nous disant : on va étudier les solutions possibles. dans mon département de l'Orne 28 pourcent de la population active est lié à la filière du cheval, donc nous sommes évidemment extrêmement attentif à sa pérennité et et il n'y a pas de doute qu'en plus, sur ce sujet, l'amendement le précise, très bien, il y a déjà eu des rapports de l'Assemblée nationale, un rapport de la Cour des comptes, tout ça, a déjà fait l'objet aussi dans cette maison d'un travail d'expertise, donc je pense que la bonne méthode, c'est de voter cet amendement de faire travailler les services cependant la navette et puis de pouvoir ce texte reviendra au Sénat avoir l'expertise de vos services, sur une base qui sera la base du vote du Sénat, voilà donc je soutiendrai cet amendement. S'il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix cette amendement 306 rectifier bis. La Commission a demandé l'avis du gouvernement et le gouvernement a émis un avis défavorable qui pour cet amendement. Qui est contre. Eh bien, il a adopté. Amendement était adopté. Nous examinons à présent l'amendement 297 rectifier c'est monsieur le comte qui va le défendre. Si on a la présidente suisse collègues selon l'article 746 du code général des impôts, le partage des biens meubles et il m'est immeuble entre copropriétaires co-héritier co-associé à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement, une taxe de publicité foncière avant la loi du 29 juillet 2011. Ce droit de partage s'est levé à 1,1 pourcent et il est depuis l'entrée en vigueur de cette loi passée à 2 5 pourcent or cette taxe représente lors d'un partage, une somme très conséquente a déboursé par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision et c'est logique échappe à beaucoup, en effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour écrire un bien souvent à crédit concernant les biens immobiliers devront le jour où il conviendra de partager c'est bien payer un impôt lié au simple fait qu'ils sont plusieurs, en être propriétaire ainsi en cas de divorce par exemple un couple possédant un actif Net de 20 de 200000 euros devra s'acquitter de la somme de 5000 euros uniquement pour protéger procéder au partage de son actif absent significatif de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s'en acquitter se maintiennent en situation d'indivision et donc dans une situation juridique confortable pour elle, il en va de même en cas de succession ou encore lors de la vente d'un immeuble acheter en indivision pour 2 concubins, cet amendement a donc pour objet de ramener le taux de droite partagent 1,5 pourcent taux auquel il était avant la loi de finances rectificative de 2011 comme vous voyez, monsieur le rapporteur monsieur Ministre il est parfois, comme le disait notre collègue de moments où l'auto, tu l'assiette, ça a été le cas dans ce cas-là, et c'est la raison pour laquelle je propose une baisse de ce taux, ce qu'il y avait dans la injustice pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer cet impôt ce nouveau taux. Merci, quel est l'avis de la commission. Je partage assez ce que notre collègue Leconte c'est vrai qu'être pénalisé sur une sortie de des divisions, avec des coûts qui ont été relevées par loi de finance éthique 10 2011 puisque le taux est passé de jusqu'à 2 5 on peut comprendre, par contre c'est vrai que on a pas eu le temps de pour expertiser, notamment devant le coût que représenterait cette amendement repasser indice à 10 pourcent peut-être également peut nous éclairer moi à titre personnel, je suis plutôt sur une sagesse, sauf si le coût est très très élevé est-ce que c'est

ces histoires de de partage effectivement le l'oedème Théo de base, on va dire c'est plutôt autour de 2 5 pourcent et donc il y a déjà un régime de faveur, entre guillemets, qui qui est prévue pour des biens qui proviennent d'une succession d'une communauté conjugale d'une indivision entre époux ou partenaires pacsés, voilà le gouvernement souhaitait en en rester là, on note que, pour une fois vous proposer de baisser une taxe. L'augmenter mais. nous, on est plutôt sur une position donc une demande de retrait, un avis défavorable et un régime de faveur dans certains cas, on ne souhaite pas voir ce taux à 1,10 maintenant, je vois bien que ce matin il y a un engouement pour

Moi ce que je vous ai dit quand quand quand je propose une méthode assez pour soutenir, c'est-à-dire que on a la chance d'avoir plusieurs clauses de rendez-vous, quand on n'a pas les éléments, ça permet de se donner quelques jours afin d'avancer maintenant si vous voulez avancer tout de suite, ça sera contre l'avis du gouvernement, mais voilà votre assemblée naturellement pleinement responsable.

et après des années. 2 lois de finances dans cet hémicycle, on a tous compris qu'il valait mieux tenir que courir, donc cela ne met pas du tout en cause, ni vos engagements niveau promesses mais simplement argument marche dans les 2 sens, c'est-à-dire nous avons plusieurs rendez-vous, donc on peut aussi voter et revoit en des rendez-vous, ceci étant, ce qu'on signale depuis ce matin et ce qui a été signalé largement leur donne réunions de commission en ce qui concerne la méthodologie, c'est aussi les conditions dans lesquelles on travaille sur cette loi de finances il y a quelques jours, les amendements du gouvernement, était à peine sec alors que nous étions en en commission, personne n'a pu les expertises et aujourd'hui on a des questions délai je pense que tout ça ravive complètement le débat autour de la méthodologie autour de la loi de finance et de la façon dont dont nous travaillons aujourd'hui aujourd'hui en en ce qui concerne ses amendements donc moi je le je soutiendrai, il est dans la ligne de l'amendement Pillet il semble aller dans. Bon sens, merci, merci, y a-t-il d'autre demande explication de vote, je n'en vois pas. Je vais mettre au voile amendement 297 rectifier un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, la liberté d'aller et de venir être est un principe fondamental aussi entre 86 et 89 pourcent de 89 euros, pardon, le montant du droit de timbre appliquée au passeport constitue un frein manifestent à cette liberté aussi cet amendement propose de le supprimer purement et simplement je vous remercie. Merci, quel est l'avis du de la Commission. je salue la constance des auteurs pour créer un débat sur le le coût du passeport et il bon il est vrai que le passeport, état, document obligatoire dès lors qu'on veut voyager en dehors de l'Union européenne dans beaucoup de pays, donc on peut se dire ça représente une sorte de taxe alors même que l'on ne peut pas voyager du Mans du Mans Adrian européenne sans sans disposer d'un passeport et le coût pour une famille à 89 euros par passeport un effet peut-être extrêmement élevé, bon, si on regarde la France est plutôt dans la moyenne européenne, du coup, des passeports, sans doute, et cela en pour jouer une partie d'argumentation, le coût du passeport à 89 euros est supérieur au prix réel de fabrication ou de fabrication par l'agence d'achat les titres sécurisés qui y a situé autour de 55 euros, mais c'est vrai que cela sert aussi à financer ce qui est par ailleurs gratuit et heureusement parce que là pour le coup, c'est totalement obligatoire, on est pas obligé de voyager en revanche d'objets dans les temps sur le sol français de disposer, avec humour, d'identité et notamment d'une carte d'identité et cette carte est délivrée gratuitement, donc il y a une sorte de péréquation le pouls du passeport et le le tout droit de timbre supérieures sans doute à ce coût de fabrication, mais l'excédent sert à financer le coût de la carte nationale identité si l'amendement est adopté, ça priverait tout simplement l'Agence nationale des titres sécurisés, la de 126 millions d'euros et ça voudrait dire qu'il faudrait retrouver recréer 126 millions d'euros de taxes de fiscalité supplémentaire par ailleurs ce qui a un coût, c'est pas juste une taxe, c'est une taxe qui relative d'une partie du coût et l'excédent sert

L'avis du gouvernement. Comment dire, un droit de timbre minoré pour les mineurs 45 euros ou même 20 euros pour les mineurs de, de, de moins de 15 ans et que il faut avoir en tête que le passeport il est valable 10 ans

prend à bras le corps, tous ces enjeux de numérisation pour pour l'État, je peux vous le dire, et d'ailleurs, et sur le le point de recruter pour faire face à toutes ces missions 80 personnels à Charleville-Mézières, donc je signale pour Marc Laménie notamment, c'est une agence qui voilà, qui qui qui est performante et encore une fois ce ce ce droit de timbre sur les passeports, il permet aussi de de faire en sorte que la CENI soit gratuite et donc voilà le gouvernement à la même position que la Commission, donc c'est-à-dire une une demande de retrait. Madame Boulet s'Peroni est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement. Je maintiens le maintenez, monsieur Karoutchi pour explication de vote. Madame la présidente, monsieur le ministre, un amendement que nous présentons avec Philippe Dominati depuis plusieurs années et je reconnais la constance de la réponse de la Commission et du gouvernement quel qu'il soit sur le fait que, effectivement, ça coûte très bien, pardon monsieur le rapporteur général lorsque vous dites : bah, c'est vrai que le le passeport ça ça devrait coûter un peu près 55 euros, bon ça paye les cartes d'identité, bah oui, mais enfin moi, quand je vais dans un commerce si si j'achète un kilo de carottes et que vous me dites que vous mettez plus cher les carottes pour que je puisse prendre les navettes gratos le le c'est pas c'est c'est pas tout à fait, bah je, je veux dire je, je comprends pas, soit on dit parce que c'est pas la même chose quand même, on dit voilà et on propose aux jeunes générations, pas moi, je vous rassure, je déteste les voyages voilà donc c'est pas le problème pour moi je vous dis simplement qu'on pousse les jeunes générations à voyager davantage avoir l'idée d'une France Monde, avoir des visions bon très bien et tout ce qu'on fait, c'est je passe sur la taxe sur les billets d'avion, mais après, c'est le coût des passeports, en en réalité, on a des politiques et on a l'action contraire on dit on voudrait que tous les Français voyagent peu nos jeunes rencontrent que qu'soit que soit Erasmus, que ce soit les autres systèmes qui soit partout dans le monde et on nous dit : ah bah oui mais le coût du passeport, état état 55 mais s'appelle d'identités de de ce qui par définition comme moi restent la bon très bien, tant mieux, mais ça n'est pas la même politique et moi je vous dis que soit on dit il faut ouvrir la France au monde, il vaut ouvrir l'esprit des Français, il faut faire en sorte que, justement, tout le monde prennent un peu conscience et on peut réduire le coût des passeports, puisque monsieur le rapporteur général, vous dites vous-même que ça coûte 55 euros ou un sous-amendement de la commission disant qu'on ramène le coup du du timbre de 87 à 55 je le vote. Madame Prima pour explication de vote. nous parlons de quelque chose qui va certainement toucher l'agence mais qui va probablement aussi touché quelque part, les collectivités territoriales, car si nous comptons beaucoup de fabrication de l'agence, on oublie un peu trop les coûts de fabrication aussi dans les collectivités territoriales, voir, or vous savez que certaines communes aujourd'hui sont le centre de la création des des titres d'identité et particulièrement des passeports sont des coûts qui sont compensées à la marge par l'État et donc j'ai peur que, par ricochet, c'est 126 millions qui pourrait manquer soit défalqué sur les dotations, donc je ne voterai pas cet amendement. Monsieur rénal pour explication de vote. Oui, ce débat curieux parce que vous vous sincèrement lorsqu'on va à l'étranger en dehors de la zone Euro,

une conclusion : on nous dit tout ce qu'il faut améliorer la procédure parlementaire, évitant tous les gens d'avoir cet amendement merci. Monsieur pu pour explication de vote. Oui merci madame le président, je suis bien évidemment très favorable à l'idée à la liberté d'aller et venir, mais je crois que ce n'est pas le bon débat, comme vient de le dire, une fois n'est pas coutume je serais d'accord avec mon collègue Claude rénal à partir du moment où on peut circuler librement dans l'Union européenne avec une carte nationale d'identité gratuite, il me semble qu'on peut payer 86 euros pour se faire faire un passeport et ce d'autant plus que rien n'est gratuit et tout a un coût et que, il me semble que ceux qui utilisent les services publics doivent y contribuer et dans le prolongement de ce qu'a dit notre collègue Prima il me semble très important d'attirer l'attention du gouvernement pour le coup sur le fait qu'il y a des transferts de charges qui sont lourdes vis-à-vis des collectivités territoriales, le passeport, ils prennent toute leur part, les pièces d'identité, ils y prennent toute leur part Les et j'y vais justement c'est exactement ça que je veux dire ma chère collègue les changements de prénom et à partir de janvier le Pacs et j'irais même jusqu'à vous proposer, pardon de à partir du 1er novembre à partir de maintenant le Pacs qui est lourd pour une collectivité comme la mienne, Angers, ça représente 4 personnes à temps plein sans aucun transfert de recettes, j'irais même jusqu'à vous proposer, à l'encontre de ce qui vous est proposé maintenant et je regrette de ne pas avoir déposé d'amendement dans ce sens d'ailleurs et ne m'interroger, du coup, sur la nécessité ou l'opportunité de créer un droit de timbre sur les Pacs et d'affecter les recettes aux collectivités territoriales qui maintenant, assure cette mission parce que, aujourd'hui, c'est une nouvelle contrainte qui pèse sur les collectivités, je sais qu'on a échangé avec plusieurs collègues de la commission des finances, sur ce point qui pèsent sur les collectivités, c'est lourd, dit sur une collectivité comme la mienne, c'est plusieurs agents à temps plein, ça permettrait de répondre à cette contrainte nouvelle et aussi la raison pour laquelle sur cet amendement, en particulier je ne je ne veulent voter, je ne le voterai pas, parce que comme je l'ai dit tout service a un coût. Monsieur Leconte pour explication de vote. Oui merci madame la présidente, pessimisme chers collègues oui 80 et quelques euros pour une personne seule, ça ne représente pas un gros coup, mais pour une famille nombreuse et là, je rappelle que la c'est pas 10 ans mais ces 5 ans, ça peut être une dépense très c'est au moment d'un déplacement, je rappelle aussi à notre collègue qui a plus que les cartes d'identité depuis 2014, malheureusement, ne sont pas reconnus dans un certain nombre de pays parce que la la valeur la la date de validité facial, n'est pas la même, le ministère de l'Intérieur reconnaît, par conséquent, il a fallu acheter enfin pour pour beaucoup de gens, même presque pour des voyages dans l'Union européenne des passeports, parce que les cartes d'identité française, quand elles sont marquées, valable jusqu'à 2014 et ben le ministère considère qu'que sont là jusqu'en 2019, mais bien entendu, les autorités étrangères ne le reconnaissent pas donc pour faire valoir son droit à voyager, il faut un passeport dans beaucoup de pays, même dans l'Union européenne et pour les familles nombreuses, ça représente quand même quelquefois des dépenses très importantes, ceci étant il est clair que contenu de ce que j'ai pu observer sur la manière dont les cartes d'identité a été délivré au cours des dernières années, il me semble que l'État ne serait pas beaucoup d'efforts si le passeport était gratuit pour le donner dans les meilleures conditions, je rappelle les délais, les rendez-vous avec lesquels avec lesquels les délais pour prendre des rendez-vous pour obtenir un passeport, je souligne, en tant que sénateur des Français d'étrangers, les difficultés qu'il y a aussi, pour quelqu'un qui habite dans le nord-est de l'Australie à aller jusqu'à Sydney et à avoir, a rendez-vous, par conséquent, si c'était gratuit, l'État ne fait pas d'effort et nous, nous aurions D des millions de Français qui n'aurait pas de titre de, de, de, de, de, de, de, de transport, par conséquent, aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver les moyens pour que l'État garantit à chaque citoyen la possibilité d'avoir dans de bons délais à titre de transport, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est encore moins qu'à l'étranger et j'espère que nous aurons des des dispositions innovantes qui perd le le permettront dans un proche avenir.

ensuite nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 167 rectifier ce monsieur Leconte. Présidente, monsieur le Ministre, collègues, je vais essayer de de défendre peut-être par l'ensemble des amendements de de de la série parce que ça serait peut-être un petit peu trop mais au moins les, les, les 4 premiers d'un coup, en tout cas pour ce que je je je je je présente là encore ça s'appuie sur un principe qui consiste à dire que si les taxes sont trop importantes, ben, parfois on les éviter, donc, en l'occurrence il y a des opérations à partir d'opération de régulariser. Ou de demandes de séjour qui ne peuvent pas se faire dans les délais, faute de moyens,

entre 55 et 70 euros en Irak en 2 en y intégrant les cartes portant mention vent et vie privée et familiale au type de l'article L 311 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les 4 les Caps les cartes délivrées au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, donc ça c'est le 167. Le 165 en fait, si vous le permettez, Madame la Présidente à moins. Oui, je vous en prime. Le 100 65 ans fait voudrait tirer les conséquences d'une d'une augmentation qui a eu lieu lorsque nous avons voté les titres pluriannuels le gouvernement dans la foulée à augmenter les taxes liées des, des, des cartes de séjour toutefois, nous constatons que, quelle que soit la durée des cartes de séjour la taxe a augmenté donc tous, nous proposons de la ramener en tenant compte de la durée de la taxe défendre 160 168 donc restreint les cartes de paiement du VISA dit de régularisation, entrée irrégulière sur le territoire, comme cela était initialement du prévue par le législateur lors de la création de cette taxe et ramène son montant à 220

touchés par cet amendement et dans l'autre, le coût de la de la taxe, enfin, l'amendement 166 propose de supprimer le paiement d'une taxe de 50 euros devant être effectués au moment même de la demande de titre de séjour, lorsque l'on demande une régularisation exceptionnelle au séjour, cette somme n'étant pas remboursable en cas de rejet de la demande, c'est une disposition qui a été introduit par la loi de finances de 2012 et qui constitue finalement un droit d'entrer dans une procédure qui n'a pas d'équivalent dans une autre procédure administrative en France, je vous remercie. ont la même orientation la même finalité soit supprimés soit réduire le niveau des taxes sur les visas, je partage ce que dit notre collègue Leconte pourrait tout à fait complet, tout à fait honnête sur cette question depuis le le PLF 2 début 2010 depuis la loi de finances initiale pour 2017 les recettes, il a dit ne sont plus affectées les recettes pour le divorce des visas ne sont plus affectés à l'office, donc c'est vrai mais ça va néanmoins dans le budget général et il est vrai que pour le budget général, il y a toujours un coup apportant notamment dans la politique d'immigration, nous avions l'autre jour le rapport en commission, chaque année, nous avons vu le rapport de de Roger Karoutchi ne l'a vu l'autre jour encore ou dans l'examen de la mission Immigration de Taman et axée avait déjà été française, hé bien on dit il faut toujours plus de moyens et c'est vrai que les dépenses ne sont pas en baisse, les besoins sont de plus en plus important, donc là, si on devait opter

beaucoup plus important qu'en France, j'ai quelques exemples en Espagne un VISA étudiant c'est 160 euros pour une année au Royaume-Uni, c'est 337 livres pour un VISA visiteurs de 2 ans etc donc la pub à tous les pays ont des systèmes de VISA payant, ça représente un coût important de traitement avec parfois pour les consulats, et donc la, la France ne fait pas exception à baisser les taxes c'est le privé de ressources,

Quel est l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements. d'un 1er titre du séjour est aussi soumis sauf pour quelques catégories mais des formations aussi induite par le C. hier une formation civique, une formation linguistique qui peut aller jusqu'à 200 heures et hé bien, cette formation est payé par l'État, donc par le contribuable, l'étranger n'a, lui, a payé que la carte de séjour, donc le fait que cette carte de séjour, voilà qui est ce droit qui soit fixé à ce niveau-là, permet à la fois de couvrir les frais de traitements mais également voilà de de participer, de contribuer en partie assez, assez frais, liés à à des formations pour l'intégration et je sais que votre assemblée, il était assez sensible, Roger Karoutchi, effectivement le le l'évoque régulièrement dans dans ses rapports, la nécessité d'avoir un véritable après emporte Serge linguistique, notamment, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que le gouvernement souhaite, comment dire, préserver les droits et montants qui sont prévues et donc émis un avis défavorable. Y a-t-il des demandes d'explications de vote, monsieur le Leconte.

340 bon, et après ils payent le type de séjour, si bien que c'est pas 300, c'est plus de 600 euros et et là je veux témoigner du fait que, effectivement, il y en a qui ne peuvent pas, parce que même si le travail.

vouloir mettre la politique de l'immigration et de l'asile juste financée par les taxes que paieraient les étrangers, enfin c'est pas sérieux, c'est une politique que nous assumons, c'est pas finalement les étrangers qui sont en France doivent pas finalement s'autofinancer, il participe au budget lorsqu'ils travaillent

troupe, que nous allons plus vite, je vais présenter en même temps mais j'incite la Commission à regardez bien dans le détail, dans la mesure où nous avons proposé un certain nombre de

est-ce que c'est normal, absolument pas. Et comment voulez-vous après que que les personnes puissent justement payer des cours de français en complément, qui sont très chers par eux-mêmes et qui sont parfois d'une meilleure qualité que ceux qui sont offerts par l'État si finalement tout va dans les taxes pour se régulariser ou avoir un titre de séjour, donc je maintiens ces amendements. évoquait effectivement revenait sur le le droit de VISA de régularisation, mais puisque vous parlez de de République et de ce que doit prendre en charge la République est-ce qu'il est normal qu'un étranger en situation irrégulière qui se met dans un process de régularisation finalement. Eh bien. Payer moins que un étranger qui lui a fait respecter les procédures, a dû, a dû s'acquitter de droite chancelleries

à donner un avis défavorable et et vraiment défavorable à cet amendement numéro 168. Y a-t-il d'autre demande explication de vote. Oui, dans Oui, dans le prolongement de de de ma réflexion sur les amendements précédent je je suis contre aussi ces amendements, en signant les attestations d'accueil dans ma collectivité et en voyant qu'il y avait un timbre de 30 euros qu'il m'est venue l'idée de de créer un timbre sur les Pacs du du même type de montant, pourquoi, parce que, et je voudrais préciser ma pensée, aller encore plus loin, cela peut paraître choquant de faire payer, mais en réalité, dans la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, compte tenu de l'engorgement de nos collectivités le choix qu'ont nos concitoyens, c'est quoi, et se voir indiquer que il n'y aura pas de Pacs avant 5 6 7 mois compte tenu de l'engorgement soit comme beaucoup de maires le conseil aux personnes qui veulent se pacser, aller vers le notaire pour qu'il a les pouvoirs de d'enregistrer et les paquets donc gagner du temps et se voir donc payer demander des honoraires de 200 à 300 euros de telle sorte qu'il me semble que si on crée un timbre et qu'on affectait les recettes aux collectivités territoriales, on pourrait sous réserve que ces recettes soient réellement affectés désengorger nos collectivités territoriales, je suis confus de revenir là-dessus, mais je voulais préciser ma pensée. Pour explication de vote. Pas vraiment une explication de vote, madame la présidente, mais c'est une réponse à Moscou est le campus, bon on entend, on entend son sujet, mais on peut pas le traiter uniquement par un angle financier Nantes de taxes si on commence à taxer les Pacs : on va taxer les mariages aussi bon ben voilà la égalité devant les taxes et les charges publiques, enfin je sais pas mais il faut retirer cette idée tout de suite. La Prima pour explication de vote oui moi je voudrais revenir sur les propos de notre. RECAP ça serait vrai cher Monsieur chers collègues si on pouvait faire des packs sont toutes les collectivités territoriales, or il tout est concentré dans les grosses collectivités territoriales qui n'en peuvent plus et qui sont obligés aujourd'hui d'embaucher pour prendre des rendez-vous parce que il y a des rendez-vous dans tous les sens et d'un projet pour faire les choses, donc je ne crois pas beaucoup malheureusement la taxe affectée parce que je sais bien que ça ne marche pas avec Bercy détesté taxes affectées de faibles rendements mais c'est un vrai sujet qu'il faut pas je pense balayé du revers de la main. S'il n'y a plus d'explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 164 actif il y a eu 2 avis défavorables qui est pour. Il est contre. il n'est pas adoptée. L'amendement 168 rectifier avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adoptée. L'amendement 168 rectifier avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adoptée. Il en va de même pour le 169 rectifier. Et nous, il en va également de même pour le 170 rectifier et ils ne sont pas adoptées. Le 166 rectifier 2 avis défavorables même vote même vote. Nous procédons à présent à l'examen du l'amendement 171 rectifier, qui n'a pas été présenté encore laisser Monsieur le comte.

que le paiement de taxes pour la délivrance d'un type de séjour son revêtement ce renouvellement ou la fourniture d'un duplicata par les conjoints de Français étaient contraires au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité, c'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement. Vous défendez également le 172 rectifier monsieur qui sont en discussion commune. C'est l'amendement qui propose d'étendre les exonérations de taxes et droits de timbres prévus à l'article L. 311 18 du 16 à à la délivrance de duplicata, rien ne justifie que des personnes étrangères victimes de violences, ne puisse bénéficier d'un duplicata gratuit, je pense que d'ailleurs, ce serait paradoxal à quelques jours de la journée internationale de mobilisation contre la violence à l'égard des femmes de maintenir cette taxe complètement discriminatoire, enfin si vous m'invitez à ça, je défends aussi l'amendement 173 qui défend la gratuité de des titres de séjour pour la délivrance et le renouvellement d'un type de séjour bénéficiaire aux bénéficiaires d'allocation adulte handicapé et de la location supplémentaire d'invalidité, je rappelle que, sur ces cas-là, si j'insiste sur tous ces amendements, c'est là, c'est, c'est c'est parce que. Ces taxes lorsqu'elles sont trop importantes, conduisent des personnes à se mettre en situation irrégulière en situation de précarité dans la mesure où elles n'ont pas toujours les moyens de. Pour rester en situation légale sur le territoire. Monsieur Leconte le 411 rectifier n'est pas défendu, quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements.

à problèmes qui veut clairement l'existence qui pourrait faire naître une discrimination, donc peut-être qu'on dans le gouvernement, et là-dessus, c'était David sagesse et tête des rectifications auxquelles il faudra procéder si, dans un instant pour reconnaître que sur le 71 y a une vraie difficulté par cohérence avec les recommandations formulées par les défenseurs des droits, le vide, c'est plutôt sur la sagesse, sous réserve, éventuellement,

délivrance gratuite de tous les duplicatas donc on encore une fois, c'est une perte de recettes et sur le ce soir, je vois les personnes vulnérables assure mais

dans la mesure où il y a un vrai problème sans doute de conformité à la décision de la du défenseur des droits et de et le monsieur Leconte souligne à juste titre, après l'éventuelle les discriminations donc on pourrait le regarder avec avec bienveillance et avis défavorables sur les autres.

Un sous-amendement parce que autant nous pouvons vous suivra pour exempter les étrangers victimes de violences conjugales et de traite des êtres humains pour l'obtention d'un duplicata du type de séjour naturellement

Je vous propose, au bénéfice du vote d'un sous-amendement par exemple du gouvernement qui supprimerait votre petit 2 dans le grand teint à ce moment-là, nous pourrions adopter votre amendement 171 qui s'. C'est. En fait, le petit train du grand c'est la proposition que je vous fais pour que nous puissions avancer dans le sens que vous souhaitez. Et par ailleurs, sur le 172 ça sera un avis favorable du gouvernement. gouvernement. Sur le 171 donc, le 172 avis défavorable. Favorable industrie favorable, très bien et 171 ça serait un avis favorable sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement. 73 Monsieur le Ministre. Alors attendez. Le 173 c'est une demande de retrait pour le coup. Voilà mais je, je trouve que, on a l'occasion de pouvoir avancer sur 171 donc je vous tends cette cette pour avancer sur le petit hein, mais on a besoin de à ce moment-là, de supprimer le petit 2. Il y a Monsieur le comte je je me permets de résumer très rapidement, le 171 rectifier. Pourrait être assorti d'un avis favorable, à condition de d'accepter un sous-amendement du gouvernement qui serait celui de supprimer le 2ème alinéa du grand temps néanmoins si vous le retirez c'est le 172 rectifier qui serait assortie d'un d'un avis favorable.

mais j'aimerais quand même comprendre parce que ce que j'ai indiqué, c'est que pour les conjoints de Français, il y avait un vrai problème aussi de discriminations

je, je, je prends déjà ce que vous nous donnez, mais le problème de discrimination pour les conjoints de Français va subsister, donc j'aimerais au moins si on avance sur ce point que vous puissiez nous dire que sur les conjoints de Français, on va travailler parce que voilà, on peut pas abandonner, surtout à partir du moment, le défenseur des droits, a aussi souligné cette cette discrimination qui était aujourd'hui en oeuvre et que vous ne proposez pas de supprimer si j'accepte votre sous-amendements, donc je prends, mais je préférerais que vous nous donniez un petit peu plus. Auteur générale. Vous allez sur le caractère un peu technique, et on a essayé d'avancer en séance pour bon si le nommant propose un sous-amendement au 171 et qu'il devait être adapté, ça revient au 172 donc la suggestion de la commission, c'est que Monsieur le comte retire le 171 et que l'on se rallie au 172 sur lequel également un avis favorable et, bien sûr, lorsque la avis favorable de la commission sur le 172. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. C'est ce que j'avais proposé monsieur monsieur Leconte, que faites-vous est-ce que vous retirez le 171. Je, je, je, je, je peux le retirer, je dirais, contraint et en même temps, repreneur étant reconnaissant de de l'avancée que cela propose je demanderai quand même Monsieur le Ministre, si il peut s'engager à ce qu'il a un travail de fait pour les conjoints de Français qui doivent aujourd'hui financer leur présence sur le territoire et c'est une discrimination qui ne peut pas subsister à long terme que vous ne souhaitait pas le faire aujourd'hui parce que vous êtes pris de cours d'accord mais on ne peut pas rester jusqu'à l'année prochaine sera l'puis on aura le même débat l'année prochaine, donc je préfère qu'on avance aussi sur ce sujet et je le retire le 171 on va voter 272 et je suis mais j'aimerais, monsieur, que vous me disiez disiez ce que vous pensez de cette discrimination pour les conjoints de Français. Monsieur le ministre est-ce que vous levez le.

Qui est contre. Il était adopté. Je mais au voile amendements sont 73 rectifier. Avec une demande de retrait du gouvernement n'avis défavorable de la commission. Y a-t-il des demandes, explications de vote qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adapté. Nous allons examiner l'article 16 ans un amendement 231 qui est présenté par Monsieur Savoldelli. merci, madame la présidente, monsieur le ministre et chers collègues, la 3 amendements qui vont évidemment s'emboîter les uns dans les autres, il s'agit. à défaut d'obtenir une augmentation de la la qui nous permettrait quand même d'annuler ce qui nous a semblé, à nous, notre groupe assez désastreuse, puisqu'il y a eu quand même 11 milliards qu'ont été prélevés sur les collectivités antérieurement à cette nouvelle majorité, je ne développerai pas pourquoi le faire pourquoi, parce que les collectivités vont être confrontés à un coût de transfert de charge provenant de l'État et qu'il faudra bien y faire face, nous avons eu l'occasion d'en parler ici, mais regardez le doublement des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire, on peut lui être unanimement favorable, néanmoins qui payent des investissements locaux. Est-ce que on peut dire que l'État assume totalement ce qui est généré, comme nouveau coup de fonctionnement. Les élus qui se qui sont là, répondront à la question, j'ai pu comprendre aussi que, sur la foi de l'expérimentation des petites classes que l'initiative serait reconduite et élargie aux autres niveaux de l'enseignement primaire. Donc ça va être un nouveau cumul de dépenses pour les collectivités territoriales en termes d'investissements aussi en termes de fonctionnement. Et s'agissant de l'école, je continue le fonds d'amorçage destiné à aider les collectivités mettent en les activités périscolaires a été ponctionné de 136 millions d'euros. Donc, si on se met dans la durée, il serait dommageable que les inégalités qu'elle soit de nature spatiale social, économie fracture encore plus la population de notre pays et touche singulièrement les enfants par une forme de traduction devant l'incapacité ou l'impossibilité pour les élus locaux de répondent par la qualité de service au défilé nous emploi du temps, d'autant que la suppression ou la compression massive des emplois aidés n'a rien aider et il est encore un domaine dans lequel l'action des collectivités locales est étroitement dépendante des effets des politiques nationales et là bon nombre d'entre nous avons une expérience au niveau du département, c'est l'ensemble du Champ social, cela commence avec le RSA, dont le coût est d'autant plus élevé que la tendance ces derniers mois est une tendance à la cristallisation de la situation des privés d'emploi avec un allongement sensible des périodes de chômage des publics les plus vulnérables, je pense aux jeunes de moins de 30 ans, où les salariés de plus de 50 ans, et cela se poursuit avec les débats toujours ouvert sur la prise en charge de la dépendance et l'autonomie des personnes âgées. D'autant que, année après année la compensation de la charge par l'État, s'avère de plus en plus déconnectés de la réalité des dépenses et qu'il faudra aux collectivités locales les moyens nécessaires pour maintenir la socialisation des plus anciens et de leur donner toute leur place dans la cité, donc, la dotation globale de fonctionnement, tels que nous souhaitons d'avoir fixé ne sera pas trop, donc c'est au bénéfice de ses observations que nous vous invitons, y compris le rapporteur général adopté cet amendement de notre groupe. Toujours dans le cadre de des 10 amendements, discussions communes l'amendement 232 c'est toujours Monsieur Savoldelli. Les départements, j'en parlais dans mon propos précédent ont quand même eu 11 pourcent de la part des gestes qui leur a été coupée, cela représente 1,1 milliard d'euros, on peut considérer que c'est considérable, il faut donc sortir les départements situation inextricable dans laquelle ils ont été enfermés et voyez, il n'y a pas d'égoïsme note pas, par exemple, j'ai beau être dans un département qui est celui du Val-de-Marne je ne fais pas partie des des départements heureusement pour ma population qui risque d'être en cessation de paiement, par contre quand je provoque d'amendements, je pense à des départements, y compris dirigés par des présidents de droite qui se retrouve en situation de cessation de paiement, voilà, donc ça c'est un autre état d'esprit, c'est pas de la posture ou de la caricature, donc cette situation, c'est de refinancer ce qui vous est proposé, c'est de refinancer des services publics de solidarité indispensable aux personnes âgées handicapées et aux personnes vulnérables ce fonds d'urgence a été annoncée, heureusement quand même, il faut lui souligné les choses quand elles sont positives, donc il y a un fond d'urgence dans une cabine reconnaissance nationale du problème, mais voyez 100 millions d'euros répartis à travers 19 départements qui sont les plus en difficulté, ne semble pas à la hauteur, nous considérons que l'urgence c'est 620 millions c'est ce que nous proposons dans cet amendement et de sanctuariser ces 620 millions d'euros supplémentaires,

là, on retourne sur un débat que nous avons ici, grâce à une niche d'un d'un autre groupe sur la question de la politique de la ville. Là, je vous rappelle l'appel de Grigny ainsi 800 élus locaux dont 100 maires qui ont lancé cet appel : on est là dans une situation, alors là, assez spectaculaire aussi puisque on vers ces larmes de crocodile sur les quartiers prioritaires sur la difficulté des populations et en même temps on coupe de 11 pourcent le budget de politique de la ville. Tout cela il faut ajouter des des crédits, des coupes dans des crédits dans des missions que Binic dont bénéficient les populations jeunes Royan, pas sur le débat frontal qui a eu sur la question des organismes HLM qui sont pourtant et on le sait, il y a ici des vecteurs de cohésion sociale. On a eu aussi un débat sur les emplois francs défendue par le président de la République qui nous semble pas être la seule réponse.

nous ne sommes pas encore sur une bataille de posture d'étiquettes ou de de clivages, des élus de toutes sensibilités défendent cette mobilisation pour les quartiers prioritaires, donc nous voulons la mettent une sorte, qu'on appellera un bouclier social dans ce projet de loi de finances 2018. En assurant une dotation de solidarité, une part de leur efficacité en les augmentant de près de 90 millions d'euros chacune donc de définir les moyens, l'ouverture d'un fonds prioritaires d'intervention de la politique de la ville, un fonds doté de 100 millions d'euros, voilà donc un bouclier social à votre disposition, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Merci sur le 239 c'est Monsieur Bocquet qui le défend. Oui, tout à fait, madame la présidente, un amendement de repli aussi en quelque sorte, mais plus centré sur le monde rural et notamment la revoyure dation du monde rural dans notre pays, soyons clairs et objectifs toutes nos campagnes ne connaissent pas aujourd'hui la la même situation, mais il est évident qu'il y a une certaine forme d'urgence à lui permettre de s'insérer pleinement dans l'espace national et de trouver leur place, leur rôle et surtout leur autonomie, la simple consultation des simulations de la réforme de la taxe habitation montre en creux la réalité de nos campagnes et la modestie des revenus, il est souvent la règle, les taux d'exonération de 90 pourcent et plus sont très fréquents et les 100 pourcent sont atteints dans plusieurs communes, ainsi, dans la Creuse, par exemple, seules 2 communes seront sous le seuil des 80 de contribuables exonérés même observation en Mayenne, département de notre ex-collègue Jean Arthuis, avec seulement 8 communes comptant plus de 20 pour 100 de contribuables à horizon 2022, la majoration de la dotation forfaitaire des communes rurales et l'un des outils dont nous pouvons nous servir pour accroître les moyens des collectivités que les dispositifs de péréquation existants ne peuvent pas parfaitement satisfaire et réfléchir également à cette distinction cette différence assez ne nette entre les communes rurales, les communes urbaines au niveau de la DGF cher c'est un thème qui est cher à l'association des maires ruraux de France que je veux rappeler soutenir ici. Merci sur le 577 Madame polluant. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur général du ministre, cet amendement vise à majorer la dotation globale de fonctionnement de 180 millions d'euros afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale à hauteur de 180 millions d'euros chacun, chacune, comme en 2016 et en 2017, contre seulement 90 millions chacune comme le propose l'article 60 du PLR que nous examinons aujourd'hui en effet, il nous paraît nécessaire de rappeler que pour les communes les plus pauvres de notre pays, qu'elles soient rurales ou urbaines ces dotations constitue la seule recette dynamique de leur budget, quand bien même leur contribution au redressement des finances publiques serait plus faible que les années précédentes, il faut souligner que ces communes continuent de pâtir de l'absence de véritable levier fiscal de la faiblesse des compensations d'exonérations d'impôts Directs locaux et du gel de la péréquation horizontales et-ce la péréquation n'a par ailleurs pas pour objectif d'être un simple mécanisme de compensation, mais bien un mécanisme de réduction des écarts de richesse entre communes riches et communes pauvres et de ce fait une péréquation verticale dynamique est nécessaire et c'est la raison pour laquelle cet amendement se propose de maintenir sa progression au même niveau qu'en 2017, il est proposé de financer la totalité de cette mesure par une majoration de l'enveloppe de la DGF, cette augmentation est gagée par un amendement, déposé à l'article 18 qui majore dotant les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ainsi aucune collectivité n'est pénalisé par cette majoration, je vous remercie.

au terme discussions entre l'État et les régions, à l'Automne 2016 compromis avait été trouvé et reposer notamment sur le partage d'un impôt national les régions françaises du modèle régional un milliard dans l'Union européenne et et consacrant suite à la création des grandes régions et au renforcement de la métropole quand même partenaire privilégié de l'État Panhard tique 16 du PLF pour 2018 revient sur ce compromis et ce rapport de l'État, matérialisée par l'adoption de l'article 140 de la de pour 2017 en supprimant accord 2008 le fonds ne soutiennent matière de économique le 4 à 52 millions d'euros et en le retirant de l'assiette de TVA qui sera alloué aux régions

mai question habituelle en cas de transfert s'est posé à combien estimez le coût de cette compétence alors l'IGF avait donné un chiffrage autour de 1 milliard vrai des évaluations extrêmement, extrêmement importante, les régions ont accepté, dans le cas d'un compromis, de limiter le montant de la compensation reçue à hauteur de 600 millions d'euros, ce qui est déjà un effort considérable ce montant devait être couvert via un fonds de soutien abondé à hauteur de 450 millions d'euros et par le dynamisme, estimé à 150 millions d'euros par an de la recette de TVA que les rejets des régions percevront à partir de 2018 aujourd'hui, donc, l'article 16 de ce projet de loi en retirant le fond développe homme économique de l'enveloppe de TVA transféré revient sur l'accord trouvé entre l'État et la région et les prive au passage et 450 millions d'euros censés compenser l'exercice d'incompétence, développement économique, le nôtre comme le précédent appel donc au respect de l'équilibre trouvé en 2017 et à la réintégration du fonds de soutien dans l'assiette de Téva transféré je dirais également que ce qui nous a déplu dans le débat à l'Assemblée nationale, c'est que l'on comparera les 450 millions d'euros au finalement 150 millions annuels donnés par la TVA, donc il y a là quelque chose qui n'est pas raisonnable puisque l'estimation préalable de l'IGF, été 2 milliards donc il faut pas simplement comparer les 450 millions à 150 millions par an où là, on pourrait penser que finalement c'est pas si mal mais bien avec le chiffrage 1er c'est par lustration de 1,6 milliard, c'est pour ça que les termes du compromis était équilibré et qu'il est anormal que la parole de l'État de se poursuivent pas ou ce ne merci, monsieur le rapporteur général, une petite seconde, il est dommage que donc la parole de l'État ne puisse pas finalement

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l'article 49 de la loi de finances initiale pour 2017 en introduisant au sein de l'assiette de TV alloués aux régions la part départementale de la dotation globale de fonctionnement de départements perçu par les collectivités unique de Martinique et de Guyane, cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance des collectivités unique de Martinique et de Guyane et de donner corps à la fusion du département de la région dans ces 2 collectivités sont issus. Merci, cher collègue, l'amendement 450 rectifier n'est pas soutenu, nous passons à l'examen du 419 toujours Monsieur patients. La loi de finances 2017 dans son article 149 consacre un changement de philosophie quant au financement de la DGF dirigeants et soit partir de 2018, c'est maintenant une enveloppe directement issu d'une fraction des recettes de TVA, qui vient financer la DGF des régions avec pour en déterminer le montant annuel un mécanisme intégrant l'évolution des recettes de TVA d'une année à l'autre, l'Avantage est évident, la TVA est une rentrée fiscale très dynamique en augmentation moyenne de 2,7 pourcent par an depuis 2009 la DGF des régions profitera de ce dynamisme pour autant, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique issu des fusions de leur département et région respective doivent assumer les charges de des échelons administratifs les déséquilibres financiers des départements ont mis la nouvelle collectivité dans une impasse financière ainsi par exemple le taux d'épargne brute de la collectivité de Guyane était de 0,3 pourcent dans son budget primitif 2016, alors comment avant la région affiche un taux d'épargne brute de 10,7 la faiblesse des recettes des anciens départements impact dramatiquement les Budgets de ces nouvelles collectivités, il est donc souhaitable que la part des prix départemental de leur DGF intègre le même système que la part régionale et profite ainsi d'une amie de la TVA, cela permettra au fil des années d'amortir le choc financier issu de cette fusion, le présent amendement vise donc à compléter la rédaction de l'article 149 de loi de finances pour 2017 en introduisant au sein de l'assiette de TVA alloués aux régions la part départementale de la dotation globale de fonctionnement Et de Guyane à cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance des collectivités unique de Martinique et de Guyane et de donner corps à la fusion du blé porte monnaie de la région dans ces 2 collectivités sont issus. Chers collègues, quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements. Je vais pas faire un incident de 2 séances mais j'aimerais savoir la présence d'une question : qu'est ce qui prévaut en droit est-ce que c'est des rouleurs papier ou les 2 à l'écran parce que j'ai beaucoup beaucoup de mal à suivre à l'écran par exemple, je vois 2 amendements 535 576 qui ont accroché sur le dos, leurs papiers et à l'écran, ils apparaissent, avec une seule barre donc c'est extrêmement difficile et la barbe de 131 a disparu de l'écran, alors que c'est celui sur lequel j'ai donné un avis donc j'aimerais que la direction des services informatiques de cette maison prévoit à des rouleurs qu'il soit lisible et conforme aux des rouleurs papier sinon on ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions, donc. Monsieur, monsieur le rapporteur général, nous allons nous en tenir aux des rouleurs papy. Je remercie de gammes de transmettre à qui de droit, sur le 231 qui n'est plus à l'écran, mais sur lesquels j'ai quand même néanmoins à donner un avis comme sur les 232 le 233 le 239 sur des amendements du groupe CRC qui ont la même finalité extrêmement sympathique auquel on pourrait souscrire avec enthousiasme, puisqu'il vise tout simplement à augmenter les la DGF alors selon les amendements, ça va de 310 millions milliards 9 d'euros, donc je pense qu'évidemment, pour être tout à fait bienveillant à l'égard de ces amendements, se dire qu'augmenter la DGF des départements d'autopartage des difficultés des communes, tout ça c'était pas dans le bon sens bon néanmoins c'est financé comment c'est financé tout simplement par une minoration du crédit impôt compétitivité du CCE, nous ne sommes pas pour la majorité à laquelle j'appartiens des fanatiques du CICE, simplement ces amendements aurait une conséquence immédiate, ça augmenterait les impôts des entreprises

n'alourdissement considérable de la fiscalité des entreprises concernant l'amendement suivant qui doit être le 577 il vise à majorité à majorer la DGF 280 millions d'euros pour augmenter la péréquation verticale. Je prends la commission a préféré donner plutôt un avis. Bienveillant soit demandant 331 qui est porté par les rapporteurs spéciaux de la mission qui sont Charles et Claude rénal cet amendement de ces 2 rapporteurs spéciaux augment déjà l'effet répartis évacuation verticale, certes dans une moindre mesure, mais. La demande de la commission, c'était une demande de retrait sinon un avis défavorable retrait au profit de l'amendement numéro 331 donc avis défavorable, demandes de retrait sur le 577 le suivant, et le 535 de de Monsieur Dantec de son groupe qui rétablit de 450 millions le foie exceptionnelle région alors c'est vrai que ce qui, d'une promesse. Du gouvernement précédent, qui avait promis aux régions de leur donner 450 millions d'euros même. Il les ressources des régions augmentent en 2018 par rapport à 2017, il apparaît néanmoins que cette promesse était une promesse de pure forme, parce qu'elle n'était pas financé budgétairement, néanmoins je vais demander aux garnements de la avis au ministre sur la position qui est a à l'égard de cette promesse et ceux qui se considèrent ou non lié par la promesse du présent gouvernement, donc avis du garnement sur l'amendement 535.

en intégrant notamment la DGF départementales pour école et de Guyane et de Martinique à la base de fractions de de la TVA a priori sur l'amendement 419 l'avis de la commission est défavorable car cela conduirait à traiter différemment des régions selon quelle forme ou non une collectivité unique en revanche le le problème soulevé par l'amendement 419 nous paraît plus pertinent et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais entend le gouvernement puisse. On voit qu'il y a bien un traitement différencié. Des collectivités ultramarines par exemple s'agissant d'outre-mer, les les collectivités le mais collègues perçoivent bien la DGF mais le montant de cette DGF et tout à fait différent de celui de la métropole, en métropole, 62 euros en moyenne bien sûr et alors que le ce montant situe plutôt autour de 20 à 40 euros concernant les régions outre-mer

qui vise à augmenter la DGF de 4 milliards d'euros effectivement nous nous approchons du mois décembre, néanmoins, vous comprendrez que le gouvernement s'en tiennent déjà à la rupture, qui consiste à stabiliser à DGF après qu'elle ait diminué, tous les ans depuis 2013, donc ça sera un un avis défavorable de façon générale, le gouvernement a les mêmes appréciations que la commission sur cette salve d'amendements sur l'amendement 232 qui vise à augmenter la la DGF au département de 590 millions d'euros il y a un dispositif qui va arriver prochainement en discussion ici, qui est dans le cas du collectif budgétaire a mise en place, effectivement, du fonds d'urgence de 100 millions d'euros par ailleurs le ministre l'a dit, des comptes publics, il était ouvert dans le cadre du travail contractuel qui va s'engager avec les 319 plus grosses collectivités à ce qu'une réflexion est lieu par rapport aux allocations individuelles de solidarité voilà doivent-elles être prises en compte ou pas dans la norme d'évolution de la dépense, on parle bien d'évolution de la dépense et pas de baisse de dépenses ce point être important et donc c'est une c'est un avis défavorable également sur l'amendement numéro 233 qui vise à augmenter la la DGF de 380 millions d'euros pour financer une augmentation, notamment de la DSU et le dessert, je voulais rappeler que, au sein de l'enveloppe de DGF qui est, je le rappelle, stabilisé dans le cas du de la copie qui vous est présenté par le gouvernement au sein de ce montant, le niveau de péréquation dans le cadre justement de la lutte contre l'inégalité territoriale et lui aussi augmenté, avec une hausse à parts égales de 180 millions d'euros pour la déçu et la DSR, qui vient après une augmentation se clef de 380 millions d'euros l'année dernière donc pour ces raisons, ce sera également un avis défavorable sur l'amendement 239 en fait, lui aussi, visé à augmenter, a déjà des départements de 500 4 à Lyon d'euros donc je m'en réfère aux propos que je viens de tenir avec du coup un avis défavorable l'amendement 577 également sur la progression de la DCRI, je vous rappelle donc on on l'augmente la péréquation cette année dans le dans le PLF d'ores et déjà, et nous souhaitons nous en tenir à ce niveau-là, donc c'est un avis défavorable défavorable pour l'amendement 560 535 et 576 les 2 amendements sur lequel la Commission souhaitait entendent le gouvernement c'est l'amendement relatif effectivement au fonds exceptionnel de soutien aux régions, qui avait été instituée par la LFI pour 2017 bah dans le mot fonds exceptionnel il y a le mois exceptionnel et et donc ça veut bien dire qu'effectivement, il n'avait pas vocation entre conduisant tant que le précédent gouvernement avait peut-être laissé entendre, avait pris des engagements, hé bien c'est vrai que si on prend le chapelet de mines, qui a été laissée par dans le précédent PLF qui a conduit d'ailleurs à prendre : apprendre à ce train de mesures de régulation budgétaire cet été,

non on va l'avenir différemment, on a le gouvernement propose d'affecter de la TVA, la TVA est une recette très dynamique de leur de plus 5 pourcent à l'heure actuelle en progression et et donc ça va permettre aux régions d'avoir 100 millions d'euros de plus par rapport au montant de DGF qu'elles avaient précédemment, donc c'est pas rien et pour donner un petit ordre d'idée, font exceptionnelle de 450 millions d'euros sur une légère qui a présenté 4 milliards d'euros pour les régions, quelles collectivités auraient ainsi plus 10 pourcent de d'attribution, j'en vois assez peu et donc je trouve que il faut valoriser assagi justement juste valeur déjà cette affectation de TVA, encore une fois, recettes, dynamique et qui produira des effets positifs de lors de plus de 100 millions d'euros dès cette année sur les amendements 418 450 et 419 présenté par Monsieur patients Karam j'entends bien, là l'appel à prendre en compte la spécificité ultramarine le 1er ministre a pu d'ailleurs à la Martinique, il y a quelques semaines, évoquer ces sujets-là, je pense qu'il faut utilement mettre à profit les états généraux des des des outre-mer pour pouvoir continuer à la réflexion, on a un petit sujet de jurisprudence parce que effectivement il pourrait y avoir si nous adoptions les amendements, l'État, cela pourrait poser la question pour d'autres collectivités qui sont en train d'être d'aller vers la collectivité unique, je pense en particulier à la Corse qui va rentrer dans ce régime, à partir du 1er janvier 2018

qui n'aient pas souhaité à ce stade et donc je souhaiterais qu'on puisse voilà, obtenir le retrait de ces amendements, sachant que, effectivement, il faut continuer à à réfléchir à la meilleure prise en compte des spécificités qui sont celles d'État et 3 ultramarin, dans le cas de l'exercice qui est conduit par Annick Girardin et et je sais que vous y contribuer ardemment voilà madame la présidente, les la position du gouvernement sur les différents amendements qui viennent d'être présentés. Oui, monsieur le ministre, sincèrement, j'ai entendu vos arguments, je les avais un petit peu pareil préalablement mais vous les avez les avez peut-être pas entendu totalement le fait que j'avais paraît un peu tous ces arguments puisque ils sont sortis à l'Assemblée nationale, on les connaissait et le fait de les répéter, donc c'est pas des arguments, juste un, on vous l'admettrez, non, moi ce qui me gêne le plus dans cette affaire. Pour l'avenir, d'ailleurs, hein, c'est je me méfie beaucoup d'humour, promesse, je trouve que quand on, gouvernement, moi j'ai tendance à dire l'État quand l'État prend des engagements par rapport à des collectivités dans un cadre négocié, on n'est pas dans une province on est sur un engagement de l'État, et moi je trouve bien que les gouvernements d'ailleurs a toujours honoré la République que les gouvernements passent en lisant après les autres, hé bien on maintienne en garde Les ses engagements, c'est tout à fait différent d'une promesse, une promesse dans un discours électoral devant de grandes assemblés, là, on comprend que ça n'engage personne mais quand à Bercy, on se réunit avec des régions, et que on signe un protocole ou qu'en tout cas on est un accord qui soit exprimés par un gouvernement, c'est pas un gouvernement, c'est l'État, et moi je pense que pour l'avenir, c'est très inquiétant dans le mot négociations, ça veut dire d'ailleurs qu'il faut arrêter toute négociation entre acteurs, un an avant les élections futures ça sert à rien d'avoir des discussions et donc ça bloque non sur 5 ans voilà donc ça fait déjà 20 pourcent de glaciation de la réflexion entre l'État et qui que ce soit, donc je pense que c'est pas raisonnables, vous pouvez dire que vous avez fait un autre choix choix pouvait dire que vous coupez pour des raisons qui vous regardent, mais cela étant dit, ce n'est pas juste et dire que les 100 millions par an de t'évader ne compensait la réponse est bien sûr non puisque elles étaient déjà intégré dès le départ par rapport à un coût coût était évalué au départ à 1 milliard 6 revues un milliard, accepté par les régions, dans le cas déjà d'une négociation à 600 millions je crois qu'on ne peut pas revenir sur l'état d'une négociation Edelstenne ailleurs ce que les régions vous ont dit, monsieur le Ministre, toutes couleurs confondues, voilà, il y a eu des accords sur le fait même que l'on puisse revenir sur n'avec l'État. Madame Prima pour explication de vote. Oui merci madame la présidente, moi je, je voudrais dire qu'il est temps de de siffler la fin de la récréation sur les collectivités territoriales et l'abondance de ses amendements le montre lorsqu'on est une collectivité territoriale on a subi, depuis maintenant 4 5 ans et mes reproches ne sont pas les reproches en réalité une constatation, mais je crois qu'il faut qu'on arrête l'application de la loi nôtre avec des conséquences sur les collectivités territoriales et la loi métropole avec des refondation de PCI, on a changé 4 fois ce qui me concerne, de territoire de PCI en 5 ans, nous avons des baisses de dotations une 1ère salve au dernier quinquennat une nouvelle salle qui nous est annoncé au prochain quinquennat des contrats de ruralité qui vont, qui viennent des réserves parlementaires qui disparaissent, des transferts de compétence de l'État vers les collectivités territoriales qui ne sont pas compensés, on nous annonce désormais la suppression de la taxe d'habitation, mais même si cette haute assemblée a eu la sagesse de d'annuler cela on a en réalité des actes de recentralisation qui sont vraiment évident, avec une perte complète de la visibilité de la prédit la prédictibilité des Budgets pour les élus locaux, en particulier donc je pense qu'il est temps d'arrêter tout ça, on nous donne des dotations les remplace par la TVA ont l'air changeons les baisses, on nous en promet on nous leur prend 6 mois après, ça devient insupportable pour les gens qui sont en charge de la véritable conduite des politiques publiques locales, donc, vraiment j'appelle de mes voeux le gouvernement pour qu'on ait enfin une trajectoire qu'on ait enfin des engagements qu'on est enfant et qu'on inscrive dans la loi une pérennité des mécanismes parce que ça devient pour nos collectivités territoriales pour les élus de la République qui serve nos concitoyens absolument insupportable.

en revanche, pour 419 je maintiens cet amendement parce qu'il s'agit de corriger une disparité qui existe entre les communes hexagonal, les collectivités hexagonal et celle d'outre-mer, cette mesure, si elle était adoptée, permettrait il y a une collectivité d'outre-mer, de gagner 5 millions 4 au lieu 2 millions 7, donc 3 millions de plus à ce qui n'est pas énorme pour le budget

On y reviendra peut-être à à doses occasions mais le rapporteur général, a été très clair et avec des propos très cohérent, puisqu'il a fait le lien entre les exonérations fiscales et les dotations de l'État aux entreprises avec les collectivités territoriales, c'est ça le mérite de la clarté.

mais attention sénateur Savoldelli, groupe communiste républicain et citoyen, vous inquiétez pas, on va avoir un grand moment, dialogue avec les collectivités territoriales mais c'est sur une enveloppe fermée Monsieur le Ministre. Alors le dialogue oui. Mais si vous me dites que vous allez ouvrir le dialogue, parce que le gouvernement entend avec les collectivités territoriales réouvrir une décision modificative, c'est un collectif budgétaire, voilà, parce que sinon, c'est bien, mais, excusez-moi pour les élus locaux, c'est de la com. On se met autour de la table, on se met autour de la table pour dialoguer, de la difficulté des communes et des départements, en particulier l'Angola ça été évoqué sur un transfert de responsabilité sur les régions mais ça enveloppe fermée. ce, il faut comprendre que chez les élus moi madame Prima je l'applaudis où j'ai un problème c'est qui qui nous différencie, ma chère collègue c'est que moi j'ai pas voté la suppression de l'ISF. J'ai pas voté le fait que, quand même, on va avoir 75 milliards d'exonérations. Aux entreprises. Non, mais quand même il y a les chiffres, les discussions qu'on a ici des fois, assure-t-elle, papiers d'identité sur sur les échelles le le CICE CIR le rapporteur général aussi une honnêteté politique une clairvoyance, il le dit, il y a un vase communicant entre les collectivités territoriales et ces 2 dispositifs je des calculs peut-être un peu simpliste mais moins 13 milliards pour les collectivités à venir, plus 12 milliards pour la suite CICE CIR. Donc voilà, moi je vous, je vous le dis, j'ai j'ai peur que ça craque sérieusement quoi j'ai évoqué la cessation département pour la cessation de paiement pour les départements, mais il y a un moment, à force de faire craquer un certain nombre de villes, on y viendra après sur d'autres exemples, les élus vont abandonner leur mandat, quel que soit leur étiquette politique. Parce qu'ils sont pas tous animés de faire carrière, etc, l'essentiel des élus sont des bénévoles dans ce pays et il y a un moment où on va avoir des problèmes de cohésion sociale sérieuse et là je pense que ça, il faut qu'on se préoccupe autrement que dire : on va dialoguer, on va dialoguer, on va dialoguer, on va dialoguer et le le le le fonds d'urgence il y a 100 millions et il y a, et ça enveloppe fermée voilà donc faut concerne ça. Merci monsieur Karoutchi pour explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, moi je voudrais revenir, je suis très gêné d'ailleurs sur les amendements sur la la capacité pour la région d'assurer le transfert de compétences, développement économique, je veux dire les choses très clairement, comme s'il s'était agi de ce transfert, j'étais moyennement favorable parce que je l'avais dit aux présidents de région, faites pas d'illusions, vous faire le transfert, la couleur de l'argent ou beaucoup plus tard donc, vous allez avoir la responsabilité et et les critiques des entreprises de l'ensemble des citoyens par rapport à cette capacité, cette compétence, développement économique, mais vous n'aurait pas les moyens, on a à l'époque estimé que globalement budgétairement ça devait faire 600 millions on a clairement dit : oh, bah on va vous faire un fonds de garantie 450 millions maintenant dit 150 millions moi là, quelle est la parole de l'État, à quoi ça sert de signer un accord, une convention avec l'État et, pardon de vous dire que pour la région Île-de-France pour ça que l'agacement est multiple, nous avions la présidente de la région et les présidents préalables de régions avaient signé un accord avec le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement Manuel Valls sur le Pass Navigo avec un concours financier évidemment un changement de gouvernement, merci le gros gros financiers tombe, il y a pas, on se tourne vers la présidente de région, lui, comment, comment Madame vous allez augmenter le prix du parce d'aller Go bah vient juste de ne pas avoir la moitié de la somme, je veux dire à un moment, la gestion des collectivités qui est qui, celle au plus proche des citoyens et doit pouvoir se faire sur des chiffres à peu près stabilisée quand l'État a dit aux régions, vous aurez 450 millions sur la compétence, développement économique, il faut que les régions et les 450 millions ça peut se négocier à la marge, réduire des 2 tiers la capacité en la matière, c'est c'est pas sérieux, ça veut dire que franchement il vaut mieux que les régions ne négocie plus le demandent plus de compétences parce que de toute manière si après, elles n'ont pas la capacité financière, ça n'a pas de sens, laissez vivre les régions

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le nombre d'amendements qui sont examinées, qu'ont été examinés, il en reste, de nombreux autres qui ont trait à cet article 16 mots montre bien la préoccupation unanime de beaucoup d'élus, d'élus, bah, je suis en particulier notre collègue du groupe CRC parler du bénévolat, de beaucoup non, nombre d'élus partage tout à fait parce que ce sont des inquiétudes légitimes et l'ampleur des des hommes en demandant : mais montre réellement ces inquiétudes légitimes alors l'article 16

en direction des collectivités territoriales, le 27 milliards d'euros, même si on a vu ces dernières années, les baisses à hauteur de 2 voire 3 milliards d'euros chaque année de la dotation globale de fonctionnement alors, Elior, savons, à la fois, commune, intercommunalité, département, région, on voit la situation variable de département à l'autre, d'une commune à l'autre et ce n'est vraiment, vraiment pas simple de l'autre côté, je dirais, on partage, on sait qu'il faut faire des économies à tous les niveaux, mais de l'autre côté les collectivités territoriales sont des donneurs d'ordre important pour l'activité du bâtiment et travaux publics on le dit même si on examine le fonctionnement ben je crois que c'est aussi la situation de chaque de chaque commune : l'échange de chaque collectivité qu'on est aussi en train de mesurer, donc à ce niveau-là, il faut rester extrêmement prudent en la matière, Jean merci. Merci, cher collègue Madame Tétu Annie. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapport général pour rester cohérent et solidaire envers mon collègue mes collègues ultra-marins ce matin je je veux quand même dire au ménisque, je suis assez stupéfait d'entendre ce que j'entends, ce matin, outre que les collectivités ultra-marins participent à l'effort de la mention avec les réductions de crédits, puisque on demandé l'effort à tout à tout mais je crois Monsieur le ministre, la question que j'aimerais vous poser quelle est vraiment la position de l'État par rapport au cours Lecter vite c'est ultra-marine journée l'occasion de revenir sur les financements au collectivités locales puisque la DGF participe bien sûr au fonctionnement de nos collectivités locales ultramarines mais la Christian que je me pose : quelle est la différence entre les collectivités locales ultramarines qui sont assujettis aux mêmes règles, qui est le fameux code général des collectivités territoriales, aussi bien sous le nom pour continuer et non palmiers et ici en France, quand aux assises des Outre-mer vous savez Monsieur le ministre, beaucoup d'un ministre des Outre-sont passés chez nous,

dans chaque, vous, elle, ne ment qui arrivent chaque venir y mettre de sa crème seul Monsieur le ministre, l'élu que je suis l'élue de terrain que je suis, je vais vous dire un truc, il y a une loi votée ici Femmes de loi égalité outre-mer où il y a plein plein plein plein de de solution a été trouvée, il suffit juste que le gouvernement aujourd'hui face la déclinaison on va encore venez nous faire rêver sous mon sous nos tropiques, vous voulez savoir vous voulez ça il faut arrêter son allié claires une bonne fois pour toutes et nous dire quelle est vraiment la place de nos collectivités au sein de la République, merci. Monsieur Dallier pour explication de vote. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, avec cette série d'amendements, il y en a à peu près pour tout le monde, les villes qui perçoivent la DSU, la dessert les départements, les régions, c'était pas suffit à démontrer que sur tous les bancs, la plupart des élus sont toujours aussi inquiets de l'avenir de nos collectivités territoriales, alors certes, il y a la promesse de jolies à la stabilisation de la DGF mais on voit bien que quand on commence à rentrer dans le détail, il y a d'abord c'est une promesse d'abord qui ne sera pas tenu pour tout le monde, par nécessité, pour les les communes, cantons et c'est normal, les communes qui ont de la population qui augmente quand on pense aux communes qui se regroupe quand on pense à l'augmentation de la bien sûr la DSR tout cela se fait violence dans une enveloppe fermée et donc il y a les collectivités qui vont voir baisser leur dotation et dotations de compensation, la desserte, enfin etc et le foncier bâti l'allergie reviendrait donc on voit bien que l'inquiétude est est est encore présente alors monsieur, mais je voudrais quand même vous interroger sur un point particulier, on sait que c'est dotations de péréquation, elle pose bien des difficultés, elles ont des critères qui sont complètement différents, je le dis souvent : on peut être attributaires de la DSU contributeurs prouve Plick et notre festive par exemple l'ce qui suffit à démontrer en Île-de-France qu'on est vraiment dans une complexité parfois aboutit à des situations qui sont un peu inexplicable, il y a un travail qui avait été engagé ici au Sénat, tout d'abord mais aussi avec l'Assemblée nationale sur une réforme de la DGF et peut-être une réforme de ces dotations de péréquation, est-ce que ce travail va être abandonné, tout comme l'idée de réformer les valeurs locatives semble abandonnée, alors même que la taxe foncière, même si un texte habitations disparaît, la taxe foncière est assis sur les valeurs locatives, donc, abandon de la réforme des valeurs locatives, est-ce que l'idée de réformer la DGF et c'est dotations de péréquation et toujours sur la table ou est-ce qu'on va passer 5 années, on en entend plus parler. Merci, s'il n'y a plus de demande, explications de vote, monsieur le Ministre, oui, je vous en prie. De 3 éléments rendent la présidente effectivement en réaction à ce qui et puis être dit monsieur Reina évoquait la parole de l'État ou les engagements d'un gouvernement tenu par un autre, oui, oui, oui, mais par exemple vous savez alors bon c'était, c'était le Parlement mais suite à un texte présenté par un gouvernement. Moi je me souviens en 2012 rayer d'un trait de plume, vous savez, une réforme de visant à traiter de la fiscalité antidélocalisation moins une majorité succédant à une autre, donc bon, je veux dire, vous le savez, l'idée c'est d'arriver naturellement tout en préservant l'esprit de discussion qui on peut avoir lieu de, de, de, de trouver des modalités les modalités effectivement sont distinctes, s'agissant de s'agissant des des ressources des régions Sophie Primas évoquait la nécessité de, de, de stabilité, effectivement, quand j'étais à la place de ces messieurs, en 2004 sur la loi, liberté, responsabilité locale, ce sont des débats déjà qu'on a eues sur l'affectation d'une part de TVA de TIPP, à l'époque, c'était la TIPP pour un certain nombre de décentralisation et donc on a un peu le sentiment effectivement, il y en a été l'un des votes encore quelques mois, d'avoir ce débat de façon très récurrente et donc, comme vous, j'appelle de mes voeux et je crois que c'est l'esprit dans lequel Gérald Herrmann à Jacqueline Gourault Gérard Collomb travaille, c'est d'arriver à poser des bases pérennes mais qui soit aussi issue justement d'un vrai dialogue d'une vraie discussion, et c'est l'idée naturellement de la logique contractuelle dans un contrat, on discute, on se met autour de la table et et on trouve des équilibres ensemble sans que ce soit d'en haut, et c'est pour ça que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que vous avez évoqué les baisses de du quinquennat précédent je vous suis, on peut pas parler de baisse de dotation alors je comprends bien qu'il y a argument rhétorique pour essayer de, de faire passer l'idée sur laquelle il y aurait des baisses de notation non il y a, il y a un travail sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, c'est pas les dotations les dotations encore, je le redis parce que à chaque fois, on a bien la dotation les dotations, elles sont stables et c'est une révolution copernicienne. Par rapport à ce qui s'est passé précédemment, bon voilà, donc je crois qu'il faut vraiment le le

bien vu ce qu'avait ce à quoi avait conduit les années précédentes en terme de dotations oui chaque année j'avais moins, moins 6 ou moins 7000 euros à chaque fois de de dotation, donc j'ai ce que c'est et, et de soins la sachez que on s'attache à vous proposer des mesures qui soient les plus pragmatique possible et s'agissant des outre-mer je pense que, naturellement, vous avez eu des processus d'assises il y a, il y a, il y a plusieurs à l'etc, mais je crois que la démarche que porte Annick Girardin en sincérité, elle est quand même très ouverte, très inclusive et que nous n'attendons que ça que de construire avec vous l'avenir des Outre-mer cesse agissant de la proposition de monsieur patients. des départements d'outre-mer et comme comme ça, je dirais les elle n'est pas. Moindre en terme de collectivité, parce que la DGF des des régions et collectivités uniques, maintenant elle est pas calculé par habitant effectivement aller calculer la résultante, vous vous souvenez de la compensation de la suppression de la part salariale de l'ATP, et donc du coup on est dans d'autres types de schémas je ne connais pas qu'il peut y avoir un un travail à conduire, je dis que il est compliqué pour le gouvernement de souscrire à une évolution des aujourd'hui voilà et donc je maintiens la demande de retrait voilà, à défaut, un avis défavorable mon regret. Bien, mes chers collègues, il n'y a plus de demande explication de vote j'ai. Propos je vais mettre aux voix l'ensemble des amendements individuellement bien sûr. L'amendement 231 et 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté l'amendement 232 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté l'amendement 233 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté l'amendement 239 avec 2 avis défavorables qui est pour. Les contrats. Il n'est pas adopté l'amendement 577 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté l'amendement 535 et le 576 identique, 2 avis défavorables qui est pour.

qui est pour. Il n'est pas adoptée et enfin l'amendement 419 avec une demande de retrait du gouvernement sinon avis défavorable, il n'est pas retiré Monsieur patients n'est-ce pas ou je le mais aux voix qui est pour. Qui est contre.

bien, il a adopté. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.